Cependant, de nombreuses questions restent en suspens. Tout d'abord, sur le fond, la circulaire du 10 juillet indique : « Afin de garantir la santé des élèves et des personnels, [ ...] le respect des règles sanitaires essentielles doit être assuré indispensable. D'ailleurs, le masque est désormais obligatoire dans tous les lieux clos accueillant du public. Mais comment des élèves de plus de 11 ans pourront-ils rester dans une même classe, ainsi qu'en extérieur, pendant plusieurs heures avec un masque ?

Qu'avez-vous prévu pour accompagner les communes, dans les territoires ruraux ? Dans les fiches techniques, vous préconisez notamment la remise d'équipements informatiques sur initiative locale. Les collectivités ayant des budgets de plus en plus contraints, quelles aides prévoyez-vous ? pour le personnel supplémentaire qui devra être déployé pour faire face à des surcharges de travail dans les missions sanitaires.

qui est en déplacement avec le Président de la République au sujet du plan Priorité jeunesse. La question que vous posez concerne principalement les indications sanitaires, qui seront travaillées

cet égard, je tiens à remercier les maires et l'ensemble des élus, qui ont travaillé sans relâche aux côtés des directeurs et directrices de l'éducation nationale et, plus largement, de tous les personnels.

Chacun recevra une réponse adaptée, aussi bien à l'école qu'au collège et au lycée. Tous les moyens seront déployés pour garantir la reprise des apprentissages sur des bases solides. Ainsi, 1,5 million d'heures supplémentaires seront utilisées en plus du temps scolaire.

ministre, vous venez d'annoncer la distribution de masques gratuits aux plus précaires et aux personnes à risque. Mais comment sera organisée la sélection ?

Le frein, c'est la perte de nos outils de production, comme l'usine de masques de Plaintel, dans mon département, fermée depuis deux ans. Un projet pérenne d'une coopérative d'intérêt collectif est mené à Grâces, toujours en Côtes-d'Armor,

Bref, monsieur le ministre, ferez-vous enfin le choix politique de la gratuité des masques pour tous, au bénéfice de la santé de nos concitoyens ? Notre pays en a les moyens ! La parole

le Président de la République a eu l'occasion de s'exprimer dans une interview télévisée sur ce sujet. Il n'y aura pas de distribution gratuite pour tous de masques, ce qu'aucun pays au monde, d'ailleurs, ne fait.

Monsieur le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, une tragédie se déroule sous les yeux du monde entier en Chine : arrestations massives et arbitraires, camps d'internement et de rééducation, viols et tortures, stérilisations forcées et avortements contraints.

sur laquelle je me suis déjà exprimé hier. Effectivement, l'ensemble des témoignages et des documents relayés par la presse

Elles vont à l'encontre des principes universels inscrits dans les grandes conventions internationales des droits de l'homme. Il est question d'internement des Ouïghours, de camps de détentions massives, de disparitions, de travail forcé, de destruction du patrimoine culturel ouïghour, en particulier des lieux de culte, de surveillance de la population et, plus globalement, de tout un système répressif mis en place dans cette région.

Nous continuerons, mesdames, messieurs les sénateurs, à condamner fermement ces pratiques. Je constate que les autorités chinoises ont réagi aujourd'hui à mes propos. Nous avons bien pris note de leur réponse. Pour autant, nous maintenons nos positions. Elles sont bien connues des autorités chinoises, puisque le Président de la République, lorsqu'il s'était rendu en Chine en novembre dernier, en avait fait part avec beaucoup de fermeté. Nous poursuivrons notre action.

Monsieur le ministre, nous prenons acte de vos déclarations, que nous approuvons. Mais nous pensons que cela ne suffit pas. La France doit agir de deux façons : au niveau européen, en engageant des sanctions économiques contre la Chine, et et à l'échelon international, en enclenchant le processus qui pourrait conduire la Chine à rendre compte, demain, de ses actes devant une juridiction internationale. Certes, nous avons des intérêts économiques avec ce pays, personne ne l'ignore.

depuis François Mitterrand en 1982 à Cancún, la France a toujours pris la défense des peuples opprimés partout sur la Terre. Aujourd'hui encore, il revient au gouvernement auquel vous appartenez et au Président de la République de se montrer à la hauteur de l'histoire, à la hauteur de notre histoire.

sont très claires : il convient d'adopter une fiscalité du numérique efficace et de moderniser la politique de la concurrence en Europe. Sur ce dernier point, les récents travaux du Sénat contiennent des recommandations pertinentes. Nous ne pouvons plus accepter que les Gafam payent des impôts dérisoires au regard de leurs profits et que la distorsion de concurrence en matière fiscale soit reine au sein de l'Union européenne

Force est de le constater, le dossier est sensible. L'échelon européen, bien que pertinent, reste semé d'embuches, dont la plus importante est certainement l'unanimité. Ayons le courage de créer, sur ce sujet, un noyau dur, qui, à terme, entraînera d'autres États. Pensons à une coopération renforcée efficace. Je me limiterai à soulever deux points primordiaux dans le cadre de la relance. Premièrement, quelles sont les prochaines étapes entrevues par la France concernant le dossier de la taxation du numérique et l'actualisation de la politique de concurrence européenne ? L'urgence est là ! Deuxièmement, à quand le début d'une harmonisation fiscale réaliste à l'échelon européen ?

Il faut apporter une réponse. Nous le savons, les règles de la fiscalité internationale ne sont pas adaptées pour mettre fin à cette distorsion. Vous l'avez dit vous-même, la meilleure réponse est internationale : telle est la position du Gouvernement.

D'autres pays tels que l'Italie, l'Espagne, l'Indonésie, ou encore la Turquie ont effectué une démarche identique et nous accompagnent dans cet effort. Pas plus tard que samedi dernier, l'OCDE a de nouveau affirmé sa volonté d'une position commune et s'est fixé l'objectif d'un accord international sur la question de la fiscalité du numérique d'ici à la fin de l'année.

Vous avez souligné avec raison le caractère historique de l'accord intervenu ce week-end lors du sommet européen. À l'occasion de la négociation de cet accord, le Président de la République l'a rappelé hier soir, la question du numérique a été posée.

a toutefois informés qu'il ne pourrait être présent. Depuis quelques semaines, les actes de violence, de nature délictuelle ou criminelle, se multiplient à l'égard de policiers, de gendarmes, de pompiers ou, tout simplement, à l'égard de nos concitoyens. Vous avez indiqué, monsieur le Premier ministre, que vous souhaitiez recréer des juges de proximité, c'est du moins ce que nous avons compris. Le garde des sceaux vient de nous dire que tel n'était pas du tout le cas : il souhaite plutôt une justice plus proche de nos concitoyens. Dont acte

Vous l'avez dit, des violences ont été commises récemment à Lyon et dans sa région. Des réponses pénales ont été apportées. Depuis la fin des mesures de confinement liées à l'état d'urgence sanitaire, ces violences,

le 14 juillet dernier. La réponse pénale a été tout aussi claire, puisque les auteurs de ces faits ont été déférés immédiatement. Un jeune majeur a été condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois fermes, avec incarcération immédiate

il y a extrême urgence à mobiliser à la fois les fonds et les personnels pour mettre en place les dispositifs permettant de mener la politique pénale que vous revendiquez et que nous pouvons largement partager.

faire très vite. La qualité de notre justice, la qualité de la réponse pénale, mais aussi de la réponse civile, déterminent, avant tout, la confiance de nos concitoyens dans notre système judiciaire. À défaut de cette confiance, nous vivrons des jours mauvais. La parole est

Elle porte sur les voyageurs arrivant par avion de l'étranger. Nous comprenons, monsieur le ministre, que les contrôles à l'arrivée soient très difficiles à mettre en oeuvre. Cependant, il existe un moyen de remédier à cette difficulté : il faut exiger la présentation d'un test négatif au départ. Le problème de la déficience des contrôles sanitaires dans les aéroports ne date pas d'aujourd'hui. Nous vous avons alerté dès le 1 avril dernier. L'affichage, la présence des services sanitaires ou une attestation sur l'honneur sont notoirement insuffisants.

Il aura fallu attendre le 17 juillet dernier pour qu'un décret prévoie la mise en quarantaine volontaire de personnes venant de l'étranger présentant des symptômes ou n'ayant pas un test négatif à la covid-19. Mais ce décret n'entrera en vigueur que dans trois jours ! Bien plus, sa portée n'est pas nationale, puisque ces mesures devront être prises par les préfets. Dans le même temps, nombre de pays n'autorisent l'accès à leur sol qu'aux seules personnes ayant présenté dans le pays de départ un test négatif, quelle que soit leur nationalité. La Chine vient de le faire. Cela évite la situation ubuesque de contrôles impossibles à l'arrivée et de quarantaines invérifiables. Pourquoi n'agissons-nous pas de même, au moins pour les voyageurs venant de pays à risque ou de pays ayant mis en oeuvre de telles mesures ? La parole

combien la recherche était un élément indissociable de notre souveraineté nationale et combien il était nécessaire de la doter de moyens budgétaires au long cours, tant elle a besoin de constance et de visibilité en termes d'engagements financiers. En ce sens, l'investissement de 25 milliards d'euros sur dix ans que prévoit ce projet de loi va dans le bon sens, comme l'augmentation significative des dotations de l'Agence nationale de la recherche

mois. Il prévoit de reconnaître l'engagement, le travail et l'ensemble des missions assurées par les chercheurs et les enseignants-chercheurs au service de la production de la connaissance et de notre société au sens large.

Ils ont besoin de temps, c'est pourquoi nous créerons des emplois supplémentaires pour accompagner les chercheurs et les enseignants-chercheurs dans tous les métiers de la recherche ; ils ont besoin de reconnaissance, c'est pourquoi nous mettrons en oeuvre une revalorisation sans précédent de l'ensemble des métiers de la recherche ; ils ont besoin de moyens, c'est pourquoi nous prévoyons, non seulement de porter le budget de l'Agence nationale de la recherche à 1 milliard d'euros, mais aussi d'ajouter 450 millions d'euros,

aéroports, les voyageurs de plusieurs avions se mélangent, sans respect des gestes barrières, sans distinction entre Français et étrangers et, surtout, sans aucun suivi. Quoi que vous nous ayez répondu, monsieur le ministre,

Le comble de l'inutilité est atteint par cette attestation sur l'honneur assurant que l'on n'a pas le covid, que personne ne réclame, alors même qu'une grande partie des malades sont asymptomatiques. Ce constat alarmant est dénoncé tous, particulièrement par les médecins hospitaliers, qui voient arriver de plus en plus de binationaux et d'étrangers contaminés n'ayant connu aucun suivi depuis leur atterrissage. Une nouvelle fois, la France prend du retard ; une nouvelle fois, elle est incapable d'instaurer, autrement que sur le papier, ce que presque tous nos voisins font : des contrôles aux frontières systématiques, pas seulement incitatifs et au bon vouloir du passager. Et ne parlons même pas des 2 000 tests PCR journaliers annoncés quand près de 20 000 voyageurs arrivent chaque jour de ces zones rouges ! Ma question est simple : allez-vous mettre en place des contrôles obligatoires et réels, afin d'éviter que nos aéroports ne deviennent des passoires à covid ? Madame la sénatrice Procaccia, il me faudrait plus de deux minutes pour répondre factuellement à votre question, ne serait-ce que pour présenter les chiffres. Vous affirmez que la dangerosité vient de l'étranger ;

nous mettons à leur disposition des tests à l'aéroport et nous les accompagnons dans une quatorzaine, le cas échéant, jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier d'un test. Croyez-moi, nous sommes déterminés sur ce sujet. Nous n'avons absolument aucune envie de permettre au virus de circuler,

de la recherche et de l'innovation, vous connaissez parfaitement l'enseignement supérieur, vous en êtes issue. Vous ne pouvez ignorer ses problèmes, vous les avez vécus. Dès lors, il est difficile de comprendre pourquoi, dès votre arrivée à la tête de ce grand ministère qui prépare l'avenir de nos jeunes, mais également de notre pays, vous n'avez pas lancé immédiatement un grand plan de relance globale sur le quinquennat, afin de rattraper les sous-investissements structurels dont souffrent nos universités. Les investissements ont été insuffisants depuis vingt ans, c'est un fait, mais c'est aujourd'hui le problème majeur. Il faudrait ouvrir une nouvelle faculté tous les ans pour accueillir les plus de 30 000 étudiants supplémentaires, alors que la dotation par étudiant ne cesse de baisser : elle est à l'heure actuelle au niveau de 2008. Ce problème financier pèse également sur l'emploi,

de plus, ces crédits, qui reposent sur des appels à projets, ne sont pas garantis. Les universités ont besoin de moyens maintenant et ne peuvent attendre le prochain quinquennat. Madame la ministre,

prévue non plus pour la mise en place, pendant l'été, d'un enseignement à distance, qui requiert pourtant des investissements, alors que vous avez refusé, ici comme à l'Assemblée nationale, tous les amendements qui tendaient à soutenir les doctorants et les boursiers pour la rentrée prochaine. Rassurez-nous, madame la ministre, en nous disant que vous avez réservé vos efforts pour le projet

pour préparer cette rentrée universitaire, avec des formations à distance. Le financement des doctorants ne serait pas assuré : nous avons prolongé d'une année la possibilité de disposer de contrats doctoraux financés

pouvoir qu'en 2017. Il nous était très difficile de construire une université par an et, surtout, de rattraper ce retard. Oui, le plan Étudiants a permis de réinjecter 1 milliard d'euros

nous aurons fait seize fois plus qu'entre 2012 et 2017. Oui, on pourrait toujours espérer plus, mais le mieux est parfois l'ennemi du bien et je préfère que nous commencions à investir sincèrement et réellement dans l'enseignement supérieur et la recherche. La parole

», affichant ainsi sa volonté de réforme. Toutefois, à la faveur d'une interview donnée au, il a amoindri les espoirs que ses premières déclarations

Ce plan va-t-il être entériné ? Va-t-on pouvoir enfin commencer les travaux ? S'agissant des aménagements de peine, le Gouvernement a-t-il décidé d'étendre le nombre de centres de semi-liberté dans les territoires où les besoins se font le plus sentir ? pour le ressort de la cour d'appel du Lot-et-Garonne et du Gers. Le Gouvernement va-t-il faire ruisseler ce budget historique à venir vers les territoires ruraux les plus fragiles ? Pour finir, a-t-il l'intention de créer ces 15 000 places de prison, comme s'y était engagé le Président de la République- même si le nombre a baissé depuis -ou plutôt

je vous prie encore d'excuser l'absence de mon collègue garde des sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a dû se rendre à Roanne, où une prise d'otages a eu lieu au centre de détention. Vous nous interrogez sur la politique que le Gouvernement entend mener s'agissant, notamment, des questions pénitentiaires. Je vous en remercie, car il s'agit effectivement d'une priorité. Vous l'avez rappelé, dans son discours de passation, Éric Dupond-Moretti est intervenu très fortement sur ce sujet. Il a effectué son premier déplacement en tant que garde des sceaux dans un établissement pénitentiaire et, à l'occasion

ont été effectués depuis le début de ce quinquennat, avec une hausse d'un quart du budget de la justice. Pour ce qui est des conditions de détention, Éric Dupond-Moretti l'a dit, nous ne pouvons nous résoudre à ce que la France, pays des droits de l'homme, soit régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme

le recours au bracelet électronique et le travail d'intérêt général comme sanction pénale ont augmenté de 20 % depuis trois ans. Nous allons poursuivre dans cette voie. Pour revenir sur la question locale, en effet, aucun territoire ne doit être oublié. oublié. Dans le Lot-et-Garonne, le quartier de semi-liberté d'Agen, que vous évoquez, dispose de dix places. Notre priorité est déjà de faire en sorte que ces places soient occupées, puisque, à ce jour, selon mes informations, deux détenus

Si rien n'est fait avant le 31 juillet, une pépite technologique française passera sous le pavillon américain, une entreprise de Gironde, Photonis, leader français de la vision nocturne sur laquelle mon collègue Olivier Cadic a déjà attiré l'attention du Gouvernement à plusieurs reprises. Teledyne, une entreprise américaine, est prête à surpayer l'achat de Photonis pour acquérir sa technologie. La transaction sera possible à partir du 31 juillet si vous ne vous y opposez pas le ministre. En effet, après vérification, l'absence de décision à cette date vaut acceptation, et non pas rejet, comme il avait été dit au Sénat. Le Gouvernement s'apprête-t-il à autoriser cette cession, avec les précautions d'usage, dont on connaît parfois la fragilité ? L'objectif ne peut pas être d'encadrer cette vente, car cela renforcerait un mouvement de fond qui fragilise la base industrielle et technologique de défense en laissant partir progressivement les PME qui la constituent. Le président Macron a déclaré vouloir ramener en France les industries nécessaires à notre indépendance, c'est très bien, mais il est tout aussi nécessaire de conserver celles qui y sont déjà celles qui y sont déjà ! Allez-vous poser votre veto à la disparition d'une société emblématique du savoir-faire technologique français et affirmer votre volonté de sauver cette branche industrielle de la défense en créant, peut-être avec Bpifrance,

Vous comprendrez que l'opération que vous décrivez, impliquant des sociétés cotées, emporte un devoir de confidentialité sur un certain nombre d'aspects qui m'empêcheront certainement d'être aussi précis que vous l'attendez.

Nous avons une décision à prendre ; elle est en cours d'instruction de manière extrêmement méticuleuse. Je veux vous indiquer que, si nous devions autoriser l'opération que vous avez décrite, nous le ferions en faisant jouer toutes les prérogatives de l'État de l'État : les prérogatives de droit, qui peuvent imposer au repreneur le maintien d'activités sensibles sur le territoire national, mais aussi des prérogatives susceptibles de nous amener à imposer au repreneur des modifications substantielles dans la gouvernance qu'il entrevoit, notamment en matière d'accès à l'information d'éventuels actionnaires étrangers, ou encore de maintien sur le territoire d'activités sensibles. C'est en prenant en compte ces deux priorités que nous travaillons, que nous examinons le dossier et que nous rendrons très vite

Monsieur le ministre, le 14 juillet dernier, le Président de la République a confirmé sa volonté de limiter le transport aérien intérieur, sans toutefois définir avec précision les contours de cette limitation. certains territoires de la République n'ont d'autre alternative que le transport aérien pour être connectés au reste du pays ; c'est le cas de mon département, les Pyrénées-Orientales. Au-delà de la question pure et simple de la suppression des lignes aériennes, se pose celle de la fréquence des rotations et de la substitution de Roissy à Orly comme aéroport d'arrivée. Comme vous le savez, il est beaucoup plus facile de rejoindre Paris en venant d'Orly que de Roissy. Enfin, il semble que la compagnie Hop ! s'apprêterait à modifier sa politique commerciale ; la liaison Paris-Perpignan, par exemple, serait supprimée. Je comprends fort bien les impératifs écologiques qui s'imposent à nous tous, mais je souhaite que vous m'indiquiez les conditions dans lesquelles, en l'absence de transports aériens réguliers, le désenclavement des territoires les plus éloignés et les plus mal desservis, notamment en matière de transport ferroviaire, pourra être assuré. Le Premier ministre a indiqué qu'il mettrait toute son énergie pour faire avancer le projet de la ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. C'est une excellente nouvelle.

Depuis le début du quinquennat, ce gouvernement a oeuvré pour désenclaver les territoires, pour assurer leur attractivité et, bien sûr, pour verdir l'ensemble des modes de transport, avec la philosophie constante de bien coordonner les modes de transport entre eux et de servir les besoins spécifiques des territoires, de leurs habitants

en faveur du ferroviaire, j'en suis d'accord, la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan est un axe structurant non seulement aux plans local et régional, mais aussi à l'échelon national. Une concertation a été menée et nous serons en mesure de faire des annonces prochainement sur les modalités

signe l'engagement de l'État pour promouvoir une offre de transport complète et garantir ainsi l'attractivité des territoires, singulièrement du vôtre. Prenons garde, monsieur le ministre, que l'aménagement des territoires ne soit une nouvelle fois la victime des décisions prises dans la capitale. Pour cela, vous le comprendrez, je fais confiance à notre Premier ministre La parole est à M. Yvon Collin, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, on le sait, dans notre pays, le tourisme est particulièrement affecté par la crise sanitaire. Aussi, les mesures annoncées lors du dernier comité interministériel du tourisme en faveur des entreprises de restauration, des cafés, de l'hôtellerie, de l'événementiel, du sport et de la culture sont vitales. Cependant, j'ai deux inquiétudes.

Aujourd'hui, elles se retrouvent dans l'incertitude financière, car elles sont prises en étau entre les demandes des clients et l'attitude des grands opérateurs d'hébergement ou de transport, qui ne leur reversent pas les acomptes. Par ailleurs, je m'inquiète aussi sur le sort des centaines de TPE et de PME des secteurs connexes au tourisme qui sont menacées de faillite, faute d'un soutien plus pointu. En effet, le tourisme, c'est aussi un ensemble de commerces liés à de petites entreprises dont la production a parfois a parfois été totalement arrêtée, faute de débouchés. C'est en particulier le cas de la confiserie française, dont l'activité dépend fortement de celle de l'événementiel ou de la L'arrêt puis le redémarrage très lent des parcs de loisirs, des fêtes foraines, le manque de touristes dans les magasins de souvenirs, ou encore la faible fréquentation des aéroports, tous ces facteurs risquent de conduire à la fermeture d'entreprises d'entreprises de confiserie emblématiques de nos savoir-faire régionaux et bien souvent fierté de notre patrimoine national. Je pense, par exemple, à la maison Pécou, dans le Tarn-et-Garonne, fondée en 1880, que connaît très bien mon collègue François Bonhomme, ici présent, et que j'associe à cette question. Cette entreprise, exportatrice de dragées dans le monde entier, est menacée également en raison de l'arrêt des cérémonies religieuses. Dans ces conditions, pensez-vous, monsieur le ministre, que le recours à l'activité partielle, l'accès au fonds de solidarité, ou encore les exonérations de charges seront suffisants pour sauver ces entreprises ? Le Gouvernement ne doit-il pas envisager des aides plus spécifiques pour sauver la confiserie française et toutes les TPE et PME connexes au tourisme ? La parole

le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État, les exonérations et reports de cotisations sociales, l'activité partielle. De plus, il a accordé la possibilité de reporter les échéances fiscales.

seront complétées par des plans de soutien d'urgence aux secteurs les plus touchés par la crise, les cafés, les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, du sport et de la culture bénéficiant, par ailleurs, de mesures renforcées prise en charge à 100 % de l'indemnité d'activité partielle jusqu'au mois de septembre, bénéfice du fonds de solidarité jusqu'à la fin de cette année, avec un accès élargi aux entreprises de ces secteurs ayant jusqu'à 20 salariés et réalisant un chiffre d'affaires allant jusqu'à 2 millions d'euros, exonérations de cotisations patronales acquittées ou reportées durant les mois de mars à juin pour les TPE et PME de ces secteurs. Cela représente une mobilisation de ressources de 43,5 milliards d'euros au total, dont 18 milliards d'euros au profit du secteur du tourisme. Le projet de loi de finances rectificative comprend également une mesure inédite d'exonération de cotisations et de contributions sociales patronales, associée à un crédit de cotisations à hauteur de 3 milliards d'euros. Cette mesure permettra notamment aux TPE-PME des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l'événementiel et du sport et aux TPE frappées d'une interdiction d'accueil de bénéficier de remises de cotisations patronales sur demande.

Préville, pour le groupe socialiste et républicain. Le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat est accablant. Les actions climatiques de la France ne sont pas à la hauteur des enjeux et des objectifs qu'elle s'est donnés. Sous couvert d'affichage environnemental, le Gouvernement va droit dans le mur. pourtant pas faute d'initiatives parlementaires ! Notre planète se meurt de notre inaction. Il s'agit non plus d'une opinion, mais d'un fait. La région arctique étouffe sous la hausse des températures. En Sibérie, c'est déjà la question du coût économique qui se pose routes détériorées, bâtiments fissurés, infrastructures liées à l'exploitation du gaz menacées et menaçantes. Nous ne voulons pas être les spectateurs résignés du dérèglement climatique. Lancée en grande pompe, la Convention citoyenne pour le climat était l'occasion de faire participer les Français à la préparation de la loi,

pour concrétiser les velléités écologiques du Gouvernement. L'effet d'annonce a une fois de plus eu raison des actes, et le virage écologique est repoussé à plus tard. Nous n'aurons donc ni changement de cap ni relance verte. Tous nos amendements issus des propositions de la Convention ont été rejetés : la baisse de la TVA sur les billets de train, la prime Climat pour éliminer les passoires thermiques, le malus sur les véhicules polluants, l'augmentation du taux de la taxe sur les dividendes. Rien n'y fait, ni les alertes de la communauté scientifique, ni la voix des urnes, ni le travail des parlementaires, ni même les propositions d'un groupe de travail citoyen que vous avez vous-même constitué : sur la social-écologie, votre gouvernement reste sourd ! Il est aussi malade de son manque d'ambition que de sa doxa libérale, peu soucieuse des conséquences environnementales. Quand et comment la loi va-t-elle entrer en résonance avec l'urgence climatique ?

Comment manger mieux avec une transition agricole qui sera soutenue par la politique agricole commune ? Comment se déplacer mieux ? Les plans de relance que nous avons déjà annoncés de la filière aéronautique et de la filière automobile nous permettent d'accélérer cette transition écologique. Alors, arrêtez les imprécations. Tous les États européens ont salué ce pacte européen. Les socialistes espagnols eux-mêmes ont dit que c'était la fin de l'Europe de l'austérité Nous sommes au rendez-vous des actes ; nous sommes au rendez-vous de cette transition écologique. Nous fermons les centrales à charbon ; nous avons mis fin aux projets EuropaCity, Notre-Dame-des-Landes et Montagne d'or. Regardez les actes ! Ce gouvernement sera au rendez-vous de la transition écologique. Angèle Préville, pour la réplique. Les actes, nous les attendons encore ! Nous sommes en train de faire l'expérience douloureuse de nos limites. Il est grand temps de nous réinterroger sur notre rôle de prédation sur la nature. On dit la disparition annoncée de l'ours polaire. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. De la beauté du monde, nous ne pouvons faire le deuil face au désastre à venir. Simplement, nous faisons de la politique avec sincérité et conviction

quel maire, quel membre des forces de l'ordre, quel enseignant n'a pas entendu parler des cartouches dites « de gaz hilarant » et constaté les innombrables cartouches usagées qui jonchent le sol de l'espace public ? L'usage de cartouches de protoxyde d'azote aux effets euphorisants, nouvelle mode pour de trop nombreux jeunes, notamment, constitue un danger pour la santé publique, comme l'ont récemment souligné

une vague de violences graves et une hausse importante des incivilités- pour utiliser ce mot pudique -trop souvent causées par l'usage de ce gaz euphorisant. Le Sénat a adopté à l'unanimité, monsieur le Premier ministre, le 11 décembre dernier, une proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote. Nous avions adopté des amendements visant à interdire la vente de cartouches de protoxyde d'azote par les sites de commerce en ligne et demandé qu'une information sur les risques avérés graves sur la santé par l'usage détourné de ce gaz soit dispensée dans les établissements scolaires.

Monsieur le sénateur, cher Jean-Pierre Grand, votre question est importante, et j'ai eu l'occasion de répondre,

La séance est reprise. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des lois a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- dix-huit voix pour, aucune voix contre -à la nomination de M. Jean-Luc Nevache à la présidence de la Commission d'accès aux documents administratifs. L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française, la région flamande et la région wallonne relative à l'aménagement de la Lys mitoyenne entre

armées est favorable à l'adoption de ce texte. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse

entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune

le 10 octobre 2019, la France et le Luxembourg ont signé à Luxembourg un avenant à la convention du 20 mars 2018 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, entré en vigueur le 19 août 2019. Cette nouvelle convention permet de renforcer les échanges économiques et les investissements entre la France et le Luxembourg, tout en s'inscrivant pleinement dans la priorité donnée par le Gouvernement à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Elle intègre notamment dans nos relations avec le Luxembourg les dispositions, issues du projet BEPS de l'OCDE de lutte contre l'érosion des bases taxables et le transfert des bénéfices. À titre d'exemple, elle contient une clause anti-abus générale contre les montages ayant un objectif principalement fiscal, et son préambule précise que son utilisation ne doit pas avoir pour effet de créer des possibilités de non-imposition. La convention de 2018 contient, par ailleurs, les normes les plus récentes en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, comme en matière d'échange de renseignements ou d'assistance au recouvrement. L'avenant proposé à votre approbation ne modifie pas l'équilibre général de la convention. Il ne modifie ni la répartition du droit d'imposer entre la France et le Luxembourg ni les dispositifs permettant de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'objet de cet avenant est de modifier les modalités d'élimination des doubles impositions pour les revenus d'emploi salariés et immobiliers provenant du Luxembourg et perçus par des personnes résidentes de France. Ces modifications concernent ainsi principalement les travailleurs frontaliers qui résident en France et exercent leur activité au Luxembourg. Les modalités d'élimination des doubles impositions pour le Luxembourg demeurent, quant à elles, inchangées. il s'agit de prendre en compte les préoccupations exprimées par les travailleurs frontaliers et leurs représentants, tant en France qu'au Luxembourg, postérieurement à l'approbation par le Parlement français de la convention du 20 mars 2018.

L'avenant prévoit ainsi que les doubles impositions sont désormais éliminées pour les revenus concernés par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, au lieu d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt étranger. Cette modification, qui répond à une forte demande des travailleurs frontaliers concernés, a vocation à maintenir le principe selon lequel les revenus d'activité immobiliers ne sont imposés que dans l'État où se déroule l'activité et où sont situés lesdits biens. Elle permet de maintenir les travailleurs frontaliers et résidents français percevant des revenus de biens immobiliers situés au Luxembourg dans une situation analogue à celle qui résultait de la convention qui était en vigueur avant le 1 janvier par le biais d'une méthode d'élimination de la double imposition dont les effets demeurent équivalents. Les dispositions de l'avenant s'appliquent aux périodes d'imposition commençant à compter du 1 janvier 2020. Tels sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention du 20 mars 2018 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune. La parole Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'objectif de cet avenant est extrêmement simple : clarifier les modalités d'élimination des doubles impositions. Vous vous souvenez que nous avions examiné au mois de décembre 2018 le projet de loi autorisant l'approbation de la nouvelle convention fiscale qui devait lier la France et le Luxembourg. La commission des finances avait alors estimé que cette convention constituait une avancée significative pour nos deux pays et qu'elle permettait de moderniser les relations entre nos deux administrations fiscales. texte tenait compte des priorités de la France et des dernières normes édictées par l'OCDE en matière d'échange d'informations et de mesures relatives à la prévention de l'érosion de la base d'imposition et au transfert des bénéfices. La convention de 2018 avait trois objectifs : éviter les doubles impositions et les doubles exonérations, accroître la sécurité juridique des opérateurs des deux pays et renforcer les moyens de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Je tiens d'emblée à vous signaler que le présent avenant ne modifie pas cet équilibre et ne revient pas sur des acquis réclamés de longue date au Luxembourg. J'entends les inquiétudes que peut susciter la modification d'accords avec un pays tel que le Luxembourg. Toutefois, le présent avenant n'est qu'une simple clarification des modalités d'élimination des doubles impositions. Ce n'est pas par avenant que nous allons régler les sujets sur lesquels nous pouvons avoir des discussions avec le Luxembourg en matière de transparence, d'optimisation ou d'évasion fiscales. L'avenant clarifie les règles d'imposition des revenus d'emploi des travailleurs frontaliers et des revenus issus de biens immobiliers situés au Luxembourg. Il est donc avant tout une modification technique. Le Luxembourg, pays de 626 000 habitants, compte, parmi sa population salariée, plus de 46 % de travailleurs non résidents. Parmi eux, plus de la moitié résident en France. Au premier trimestre de cette année, il y avait plus de 107 000 travailleurs frontaliers français. Ce sont ces derniers qui ont alerté les autorités sur les conséquences de la modification des règles relatives à l'élimination des doubles impositions, à l'article 22 de la convention de 2018. Tel qu'il est rédigé, cet article laisse entendre que, selon la situation, les revenus d'emploi des travailleurs frontaliers peuvent être imposés deux fois. Selon la convention, ils ne sont pourtant imposables que dans l'État où est exercée l'activité. Or la France a choisi de recourir, pour une partie des revenus ciblés par la convention, à la méthode de l'imputation. Cela revient, pour l'administration fiscale et dans certaines situations, à imputer sur le montant de l'impôt théoriquement dû en France un crédit d'impôt dont le montant est égal à l'impôt effectivement acquitté au Luxembourg. L'article 22 laisse ainsi ouverte la possibilité pour la France d'imposer le différentiel entre l'impôt acquitté par les travailleurs frontaliers sur leurs revenus d'emploi au Luxembourg et l'impôt qu'ils auraient payé en France qu'ils auraient payé en France sur ces mêmes revenus en appliquant les dispositions du code général des impôts. Ce n'est donc pas à proprement parler un risque de double imposition, mais un risque d'une imposition en deux temps. Cette inquiétude s'est trouvée renforcée par l'adoption en 2017 au Luxembourg d'une réforme de l'impôt sur le revenu favorable, par rapport au système français, aux personnes dont le revenu est inférieur à 36 000 euros par part. Le risque d'un différentiel d'impôt entre la France et le Luxembourg était donc d'autant plus élevé. Par ailleurs, le Luxembourg réfléchit à une nouvelle réforme de l'impôt sur le revenu qui soit plus favorable aux célibataires, ce qui aurait encore plus renforcé le risque d'une double imposition. Dans le système antérieur, celui de la convention de 1958, la France avait choisi la méthode de l'exemption : si les revenus d'emploi étaient imposables au Luxembourg, alors ils étaient totalement exonérés d'impôt en France. Toutefois, l'administration fiscale pouvait en tenir compte pour calculer le taux effectif d'impôt sur l'ensemble des revenus du ménage. C'est le principe dit de l'imposition partagée, et c'est celui qui était également retenu pour les revenus issus de biens immobiliers situés au Luxembourg. La méthode retenue pour les revenus immobiliers dans la convention de 2018 a suscité les mêmes réticences que celle qui concerne les revenus d'emploi des travailleurs frontaliers. Comme pour ces derniers, les revenus immobiliers ne sont pourtant imposables que dans l'État où se situent les biens. Dans ce cadre, que fait le présent avenant, signé à peine plus d'un an après l'adoption de la nouvelle convention fiscale entre la France et le Luxembourg ? Il revient au système antérieur pour les revenus des travailleurs frontaliers et pour les revenus immobiliers et, surtout, il clarifie l'ensemble des règles relatives à l'élimination des doubles impositions. Concrètement, les revenus d'emploi des travailleurs frontaliers seront exonérés d'impôt en France s'ils ont bien été soumis à l'impôt au Luxembourg. Les revenus issus des biens immobiliers situés au Luxembourg seront exonérés d'impôt en France, mais l'administration fiscale les prendra en compte pour déterminer le taux effectif d'imposition de l'ensemble des revenus immobiliers du ménage. L'avenant entend ainsi lever toute ambiguïté et s'assurer que les revenus d'emploi et certains revenus immobiliers ne soient pas imposés deux fois. Je me répète, ces nouvelles méthodes de calcul ne créent pas d'avantage particulier : elles reprennent des dispositions que la France a déjà conclues dans le cadre de conventions fiscales signées avec d'autres pays et qui étaient en vigueur avant l'adoption de la nouvelle convention.

L'incidence sur les recettes fiscales françaises est par conséquent nulle et les acquis de la convention de 2018, qui visaient notamment à éliminer tout risque de double exonération, sont maintenus. pour revenir sur un sujet qui a été abordé en commission par Jean-François Husson, je précise que, en vertu des règles figurant dans la convention, la détermination des règles d'imposition ne se fait pas au choix du contribuable. Elle dépend du type de revenus et du lieu d'émission et de perception de ces revenus. Par ailleurs, le principe de l'imposition partagée permet de tenir compte du niveau des revenus dont l'imposition revient au Luxembourg, pour calculer le taux effectif de l'impôt dû en France. Quant aux compensations, dont je sais que c'est un enjeu majeur pour les territoires frontaliers, elles ne peuvent pas se régler dans le cadre de ces avenants et conventions.

commise en 2018 et on ne peut pas traiter les autres sujets. Malgré tout, je vais vous parler de ces autres sujets, parce qu'ils sont importants. Cet avenant,

c'est un sénateur qui vous parle -, les territoires frontaliers sont progressivement asséchés de leur tissu économique et nos collectivités n'ont plus les ressources suffisantes pour financer les nombreux services demandés par les travailleurs frontaliers. J'aborde maintenant un autre point.

équilibrées et justes. Après tout, la métropole luxembourgeoise n'est autre que la troisième métropole de la Lorraine, pour reprendre les termes du nouveau maire de Nancy, Mathieu Klein. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est la troisième fois en cinq ans que le Parlement examine une convention fiscale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg. En décembre 2015 a été ratifié le quatrième et dernier avenant à l'ancienne convention, dont la première version remontait à 1958. Plus récemment, fin 2018, le Sénat ratifiait cette fois-ci la nouvelle convention bilatérale, établie à partir du modèle standard de l'OCDE, également ratifié par la France la même année, et qui s'impose désormais à l'ensemble de nos conventions fiscales. Dans la mesure où le présent avenant, signé le 10 octobre 2019, contient lui aussi des dispositions de nature législative, il nécessite une approbation par le Parlement au titre de l'article 53 de la Constitution, un projet de loi spécifique. La nouvelle convention fiscale avait été ratifiée par le Sénat le 17 décembre 2018. Déjà, la procédure normale avait été rétablie en lieu et place d'un examen en procédure simplifiée. Tout en saluant le nouvel accord, qui visait à la fois à moderniser notre droit pour prendre en compte les standards internationaux et à mettre un terme aux pratiques passées d'optimisation fiscale, j'avais déjà signalé à l'époque l'angle mort que constituait, à mes yeux, la situation des travailleurs frontaliers, pour lesquels le nouveau texte aurait pu avoir des conséquences imprévues et défavorables. J'avais également regretté le caractère succinct de l'étude d'impact d'alors. Rappelons qu'il n'est pas possible d'amender un projet de loi de ratification : le Parlement ne peut qu'approuver ou rejeter en bloc ce qui a déjà été négocié et signé en amont. C'est la règle pour tous les traités internationaux. Ni la convention de 2018 ni cet avenant n'y font exception. La convention, entrée en vigueur cette année, établit le principe de l'imposition en France de l'ensemble des revenus perçus au Luxembourg, afin d'éviter les doubles exonérations. Mais, en même temps, les salariés résidant en France bénéficient d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt déjà acquitté au Luxembourg, ce qui empêche les doubles impositions, mais n'exclut pas une possible surimposition en France, notamment pour les plus bas salaires.

On ne peut donc qu'y être favorable, d'autant que cela concerne en particulier les plus bas salaires. On peut simplement regretter l'absence d'évolution de l'accord en ce qui concerne le télétravail, avec la question sensible du seuil des vingt-neuf jours, qui vient d'être évoquée. En cas de dépassement de ce seuil, le frontalier passe à l'imposition en France pour les journées télétravaillées, mais reste également imposable au Luxembourg. La façon dont sera effectué le décompte reste à trancher

consensus. Les grands groupes d'audit luxembourgeois, durant leurs séances d'information, précisent aux entreprises luxembourgeoises que, en cas de dépassement du seuil des vingt-neuf jours, elles doivent s'enregistrer en France pour s'acquitter de leur impôt. Selon nos informations, cela ne devrait pas être obligatoire si l'entreprise ne dispose pas de salarié soumis au système de sécurité sociale français.

Sur ce dossier, le centre de ressources Frontaliers Grand-Est mis en place par la région peut être un relais d'information efficace. Au-delà des questions techniques de fiscalité, nous devons garder à l'esprit les préoccupations quotidiennes des frontaliers les nuisances liées à l'engorgement des voies de communication, les embouteillages, la perte de temps, ainsi que les risques d'accident et la pollution qui ont des conséquences sanitaires et financières somme toute importantes. À ces difficultés, le télétravail apporte des solutions pratiques, que l'on a pu particulièrement observer pendant la période de confinement. mettre en place le cadre juridique adapté et pleinement satisfaisant pour toutes les parties. L'accord temporaire, qui a été rappelé par la secrétaire d'État Christelle Dubos à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, et qui est prorogé jusqu'au 31 août 2020, ouvre une voie intéressante. le Grand-Duché constitue un pôle économique majeur dans la région et reste un partenaire important à l'échelon européen du fait de sa situation géographique et historique. Sa position intermédiaire entre pays du Nord et pays du Sud lors des récentes négociations sur le plan de relance européen en témoigne encore une fois.

le débat -d'une véritable agglomération transfrontalière, dynamique et équilibrée. Les accords fiscaux doivent favoriser une coopération plus transparente et plus fluide entre les administrations des deux pays, tout en préservant les spécificités nationales.

Luxembourg, entrée en vigueur le 19 août 2019 et applicable depuis le 1janvier dernier, il nous est demandé d'autoriser l'approbation d'un avenant à cette convention. La convention franco-luxembourgeoise, signée en mars 2018, consistait en une mise à jour importante de la convention du 1 avril 1958, l'une des plus anciennes conventions fiscales bilatérales signées par la France. En 2018, il s'agissait surtout de tirer les conséquences des avancées obtenues au niveau multilatéral grâce à l'accord trouvé au sein de l'OCDE autour du projet BEPS.

La convention de 2018 visait à apporter deux autres correctifs notables. En matière immobilière, d'abord, elle a modifié certaines règles qui accordaient des avantages injustifiés aux investisseurs luxembourgeois. En matière de double imposition, ensuite, elle prévoyait que les revenus d'un résident français imposable au Luxembourg soient imposés en France, déduction faite du montant de l'impôt payé au Luxembourg, une mesure alors présentée comme inédite.

La méthode d'imposition par imputation retenue en 2018 prévoit l'octroi par l'administration fiscale française d'un crédit d'impôt, qui est égal à l'impôt luxembourgeois, mais qui est plafonné au montant de l'impôt français. Les travailleurs frontaliers sont donc redevables d'un impôt sur le revenu de leur travail luxembourgeois d'abord au Luxembourg puis, en complément en France si le montant de l'impôt français est plus élevé. L'avenant que nous devons approuver revient à la méthode d'imposition antérieure, qui résulte de la convention de 1958. Celle-ci prévoit que les revenus d'activité sont imposés dans l'État où se déroule l'activité. Les doubles impositions seront désormais éliminées grâce à l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant aux revenus luxembourgeois. Mes chers collègues, au-delà des points techniques exposés par le rapporteur, il faut remettre cette convention, ainsi que l'ensemble des conventions fiscales bilatérales signées avec des partenaires européens dans le contexte de la construction européenne. Cette convention, comme nous l'avions dit l'an dernier, constituait une avancée en ce qu'elle intégrait les nouvelles dispositions BEPS de l'OCDE. Néanmoins, les vrais sujets européens sont la concurrence et l'harmonisation fiscale. L'Union européenne a réussi l'harmonisation de la fiscalité indirecte, mais la règle de l'unanimité qui prévaut en matière fiscale au sein du Conseil européen est un frein. Nous connaissons les régimes fiscaux favorables de certains de nos partenaires européens. Pour l'impôt sur les sociétés, le projet européen doit être rapidement mis en oeuvre. Il devra être complété pour répondre à la question de la concurrence fiscale, soit sous la forme d'une interprétation uniforme des règles en matière d'assiette commune, soit par la mise en place de taux minimum et maximum d'imposition sur les sociétés. En conclusion, mon groupe votera sans réserve pour ce projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale entre la France et le Luxembourg, mais restera attentif aux efforts du Gouvernement pour parvenir à un accord à l'échelon européen en matière d'harmonisation fiscale. La

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur l'initiative collègue Éric Bocquet et à la demande du groupe CRCE, nous examinons aujourd'hui l'avenant à la convention fiscale entre notre pays et le Luxembourg,

affiché était de mieux lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscales : elle comporte notamment une clause anti-abus générale contre les montages ayant un objectif principalement fiscal.

pays fondateur du marché commun et de l'Union européenne, présente quelques caractéristiques fiscales qui méritent que l'on s'y attarde. C'est vrai ! Citons, d'abord, l'existence au Luxembourg de ports francs, espèces de bunkers surprotégés, inaccessibles sauf aux initiés, où sont stockées des oeuvres d'art à la valeur vertigineuse. Sacha Guitry, grand amateur d'art, aimait dire qu'il existait deux types de collectionneurs : les collectionneurs « vitrine » et les collectionneurs « placard ». Avec les ports francs, on est plutôt dans la seconde catégorie. L'anonymat des propriétaires est la règle. Nombreux sont les clients des ports francs qui créent une société offshore domiciliée dans les îles Vierges britanniques ou dans toute autre juridiction de ce type, et louent un box sous le nom de cette compagnie. Il faut également noter que le Luxembourg a fait l'objet de poursuites judiciaires de la part de la Commission européenne, pas plus tard qu'au mois de mai dernier au sujet des lois visant à empêcher le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. l'Union européenne a pris de nouvelles dispositions ayant pour but de contrôler les actifs financiers de responsables politiques et d'entreprises. Or il se trouve que le Luxembourg fait partie des États membres qui n'ont pas encore complètement mis en oeuvre L'exécutif européen a instamment demandé au Grand-Duché de modifier une loi permettant aux entreprises de réduire leurs charges fiscales au-delà de ce qui est autorisé dans le cadre des règles de l'Union, dans la mesure où cela réduit les ressources fiscales dans les autres États membres. Le Luxembourg est un pays de 600 000 habitants qui accueille autant d'investissements directs à l'étranger que les États-Unis et beaucoup plus que la Chine, indication donnée par un rapport du FMI l'an dernier. La valeur de ces investissements atteindrait 4 000 milliards de dollars. Une très grosse partie de cet argent est stockée dans des coquilles vides créées par des multinationales, sans activité réelle au Luxembourg, des véhicules financiers spécifiques, dont la seule raison d'être est de bénéficier d'une fiscalité plus clémente.

s'agit là encore d'une histoire de montages financiers complexes, impliquant des sociétés-écrans et d'autres coquilles vides, qui s'imbriquent les unes dans les autres. L'opacité de ces structures offre à leurs promoteurs une source d'enrichissement défiant l'entendement du citoyen ordinaire.

nos impôts financent ainsi des structures à l'opacité redoutable. Eh oui ! Mes chers collègues, chacun comprendra que, dans ces conditions, et au vu de ces éléments, mon groupe ne peut s'en tenir à l'examen d'un avenant. Il exprime son plus grand scepticisme quant à la valeur d'un engagement du Luxembourg au bas d'une convention fiscale bilatérale. Ce débat est une nouvelle occasion de poser des questions sur la politique de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales de notre pays et de l'Union européenne

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous pouvons nous satisfaire de débattre aujourd'hui d'un projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à une convention fiscale entre la France et le Luxembourg. Ces textes visent à renforcer la coopération fiscale entre les deux pays avec pour objectif d'éviter les doubles impositions et de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales. La négociation de la convention a été l'occasion d'un dialogue fructueux avec le Grand-Duché, au cours duquel nos deux pays sont parvenus à des solutions de compromis au service de l'intérêt commun. Les dispositions dont il est question concernent un peu plus de 100 000 Français, qui représentent près du quart des salariés travaillant au Luxembourg. Il est important de sécuriser leur situation, afin de ne pas nuire à la mobilité des travailleurs, tout en garantissant une imposition juste : ni double imposition ni évasion. Les administrations fiscales ont encore du mal à faire face aux conséquences du marché commun, sur les questions tant de fraude que de double imposition. C'est tout l'intérêt d'améliorer la coopération en la matière, afin de favoriser une fiscalité au plus près d'une réalité partagée entre deux territoires. La problématique de la fiscalité transfrontalière se pose avec d'autant plus de force au Luxembourg que près de la moitié des salariés qui y travaillent ne sont pas résidents fiscaux de cet État. Elle souligne aussi, plus généralement, la difficile conciliation dans la pratique entre, d'une part, la liberté de circulation des personnes en Europe et, d'autre part, des fiscalités encore largement nationales.

Cela permettrait à la fois de mieux identifier la fraude et de mieux la combattre. Cela serait aussi un réel progrès pour les acteurs européens et dynamiserait l'activité dans tous les territoires. L'Europe avance cependant difficilement vers l'harmonisation fiscale, dans la mesure où l'adoption de règles européennes en la matière reste conditionnée à l'accord unanime des États membres. Nous avons pu voir ces derniers jours qu'obtenir l'accord des Vingt-Sept n'est pas chose facile, même lorsque l'avenir de l'Union est en jeu. À cet égard, les pays qui souhaitent progresser sur ces sujets doivent pouvoir le faire sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'unanimité. Une Europe à plusieurs vitesses peut parfois la solution en ce qu'elle permet de faire émerger les meilleurs dispositifs et,, d'achever de convaincre ceux qui hésitaient encore. L'avenant à la convention, dont il est aujourd'hui question, est l'exemple d'une coopération qui fonctionne. Elle est fondée sur l'intérêt mutuel des États signataires et, lorsque la pratique révèle que c'est nécessaire, elle est révisée. Nous avons besoin d'une Europe qui ne craigne pas d'aller vers plus de coopération. L'euro et l'espace Schengen constituent deux forces majeures de l'Union.

en mars 2018. Certains considèrent encore le Luxembourg comme un paradis fiscal. Certes, ce pays constitue la première place financière de la zone euro et concentre les plus grands fonds d'investissement et les sièges sociaux de banques, et ce avec 600 000 habitants Effectivement, jusqu'à il y a quelques années, le système financier luxembourgeois était très opaque et s'affranchissait des règles de l'OCDE. Il y a six ans encore, le scandale des LuxLeaks avait mis en lumière certaines pratiques d'évitement fiscal. Pour autant, des progrès ont été accomplis depuis. En juin 2018, le Luxembourg- comme la France d'ailleurs -a signé une convention multilatérale tenant compte des avancées obtenues dans le cadre des travaux BEPS, menés depuis 2013 au sein de l'OCDE. Justement, la convention bilatérale dont nous discutons cet après-midi s'articule avec cette convention multilatérale. Il me semble essentiel de revenir sur l'importance du travail frontalier.

nous avons sollicité, les uns et les autres, des mesures de contrôle à titre préventif avant d'octroyer des prêts ou des garanties de l'État. Le ministre, votre collègue Olivier Dussopt, nous a expliqué à de nombreuses reprises qu'il ne voulait pas de contrôle.

-l'importance de la coopération transfrontalière entre pays voisins. La conférence intergouvernementale que certains d'entre vous ont mentionnée offre évidemment un cadre

le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (texte de la

constituant l'ensemble du projet de loi. L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2019

le rappelle d'emblée, le cap reste le même pour nous : sincérité budgétaire, responsabilité et confiance étaient les trois piliers de 2019 ; ce sont ceux de 2020 ; ce seront ceux de 2021

J'ai entendu, ici même, au Sénat, mais également parmi certains groupes à l'Assemblée nationale, des réserves et inquiétudes sur lesquelles je souhaite revenir. Tout d'abord, certains nous reprochent de mener une politique de rigueur, voire d'austérité.

; renforcement des moyens de nos forces armées et de sécurité- à titre d'exemple, les dépenses de la mission « Défense » ont augmenté de 4,4 % par rapport à 2018, à la suite de l'ouverture de crédits additionnels de 1,7 milliard d'euros dans le cadre de

: le plan d'investissement dans les compétences, qui vise à former un million de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés et un million de jeunes éloignés du marché du travail, représente un effort budgétaire sans précédent de plus de 13 milliards d'euros sur la période couvrant

J'en profite d'ailleurs, alors que commenceront prochainement les débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour faire un rappel : toujours au titre de cet exercice 2019, mais aussi dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2020,

Je souhaite rappeler que nous avons réalisé 1 milliard d'euros d'économie sur les dépenses pilotables de l'État au cours de l'exercice 2019, par rapport à ce qui était inscrit dans la loi de finances initiale. Depuis le début du quinquennat, nous avons amélioré le solde public. Le déficit est passé de 2,9 % du

Toutefois, dès l'an prochain, nous amorcerons le retour à une trajectoire de maîtrise de l'endettement et de responsabilité budgétaire, en concevant un plan de relance ciblé sur deux ans, fait de dépenses réversibles, et en maîtrisant l'évolution de la dépense pour ce qui concerne les budgets que je qualifierai d'« ordinaires

avec les responsables de programme, la direction du budget et la direction générale des finances publiques. La qualité de l'exécution budgétaire a d'ailleurs été soulignée par M. le rapporteur général en commission, et je l'en remercie. remercie. Comme en 2018, le Gouvernement n'a procédé à aucune ouverture ou annulation de crédits par décret d'avance. Les autorisations parlementaires ont été respectées et nous avons procédé à l'ajustement des prévisions budgétaires au plus près des évolutions,

Cette gestion maîtrisée s'est traduite par la baisse du niveau de mise en réserve de 8 % en 2017 à 3 % en 2019. Nous avons ainsi fait en sorte que les responsables du déploiement des politiques publiques sur le terrain puissent connaître, dès le début d'année, la réalité et la totalité des moyens dont ils disposent, puissent les engager de la manière la plus sereine, la plus autonome et la plus libre possible. C'est ce qui justifie cette baisse du taux de mise en réserve.

commencer à redresser la situation structurelle des comptes publics. C'est à ce titre, principalement, que le Sénat a décidé de ne pas adopter ce projet de loi de règlement

conduite par la majorité, à un moment où un grand nombre d'indicateurs macroéconomiques étaient encore au beau fixe. Contrairement à ce qui a pu être dit, monsieur le ministre, les chiffres ne sont pas bons pour 2019 ! Malgré une croissance

au cours de la première lecture. Ce projet de loi de règlement des comptes de l'État de 2019 est désormais, comme nous l'avons dit, issu d'un autre monde, au regard de la situation inédite dans laquelle nous sommes plongés depuis l'émergence du virus situation face à laquelle nous devons continuer de suivre des mesures strictes de sécurité sanitaire, comme le port du masque dans les lieux clos. Les propos nuancés et rassurants que l'on pouvait tenir l'an dernier quant aux perspectives de rééquilibrage et de redressement progressif des finances publiques ne sont hélas plus de mise. Depuis la fin de mars dernier, l'Insee publie des points de conjoncture à échéances rapprochées, toutes les deux à trois semaines. Le dernier point, publié le 8 juillet, a confirmé une chute d'activité de 17 % au deuxième trimestre de cette année, au lieu des 20 % précédemment estimés.

avec une certaine impatience- pour ne pas dire une certaine inquiétude -le prochain point de conjoncture, qui doit être publié avant la fin du mois. La principale bonne nouvelle du projet de loi de règlement est le déficit finalement contenu à 3 % en 2019. Si c'est hauteur de 17 milliards d'euros prises pendant le mouvement des « gilets jaunes », en particulier la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, avaient fait craindre un nouveau dérapage des finances publiques., le solde 2019 est donc relativement fidèle à la loi de programmation de 2017, ce qui mérite d'être souligné. De même, l'endettement s'était stabilisé autour de 98 % du PIB, et, pour la première fois depuis longtemps, on a constaté une baisse de la part de la dépense publique dans la richesse nationale, Ces bons résultats sont dus en partie aux recettes perçues grâce aux fameuses primes d'émission sur la dette, dont j'ai parlé en détail en première lecture. Certes, la réduction du déficit structurel aurait dû être plus importante. Il faut dire que le pilotage des dépenses de l'État est d'une extrême complexité et pas toujours d'une grande lisibilité, compte tenu des masses financières en jeu et de la multiplicité des administrations. Par rapport au budget initial, certains crédits ont été revus à la hausse, comme ceux alloués à l'aide publique au développement, en hausse de 1 milliard d'euros,

les grands périmètres budgétaires de l'État évoluent peu, ce qui traduit peut-être une difficulté à redéfinir, rationaliser et redéployer certaines de ses missions.

Toutefois, la maîtrise des dépenses s'est améliorée, grâce à des économies de gestion de l'ordre de 1 milliard d'euros. Cette bonne gestion permet d'afficher un déficit public à seulement, si je puis dire, 92,7 milliards d'euros, soit 15 milliards de mieux que dans la loi de finances initiale. peut-être été encore plus faible sans le basculement complet du CICE en baisse de cotisations sociales. Les objectifs de performance instaurés par la LOLF semblent atteints dans 50 % à 60 % des cas, ce qui est difficile à interpréter à souligner la bonne tenue des comptes des collectivités territoriales. Depuis 2018, elles ont pleinement joué le jeu de la contractualisation et contenu leurs dépenses de fonctionnement. Elles ont joué un rôle essentiel d'acteurs de proximité dans la crise sanitaire, en commandant et en assurant l'approvisionnement

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est vrai que le chaînage vertueux voulu par les concepteurs de la LOLF

cette époque paraît désormais lointaine : c'était le monde d'avant la crise sanitaire- autant dire, d'un point de vue budgétaire, la préhistoire.

que d'aucuns appellent la politique de l'offre, était déjà dans la stratégie budgétaire du Gouvernement. Il doit être maintenu, car, on le sait, la relance passera par le soutien

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous discutons à nouveau du projet de loi de règlement et d'approbation des comptes de l'année 2019. Si l'exercice relève de la mécanique parlementaire habituelle, il peut aussi nourrir le débat politique, si l'on en a le goût.

2019 n'a pas fait exception, et l'avenir n'est guère plus glorieux : le Président de la République a artificiellement renouvelé l'équipage, tout en gardant le même cap. Alors même que le pays étouffe, l'exécutif continue de pressurer les moyens de l'État et des collectivités territoriales, détériorant inévitablement les services publics. les choix opérés dégradent dans le long terme les finances publiques, puisque le Gouvernement multiplie les cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises. Un exemple : alors que la France compte environ 500 niches fiscales,

La stratégie est mauvaise, car le raisonnement à son origine est, je vous le dis, dépassé. Les exigences de justice fiscale, d'écologie, d'un État plus juste, protecteur et égalitaire sont vues, à travers l'oeillère macroniste, comme contre-productives et toujours coûteuses. Nous essayons pourtant, en relayant ces demandes des citoyennes et des citoyens, de faire comprendre qu'il ne s'agit pas de concurrence guerrière ou de rationalisation, mais de solidarité,

alors même que des mesures comme le rétablissement d'un impôt sur les fortunes ou la plus forte taxation des dividendes font de plus en plus consensus ... De petites erreurs à la marge sont corrigées, de-ci de-là.

mal an, 183 personnes sont devenues millionnaires, ce qui représente une hausse de 11 %. La France se place ainsi au cinquième rang du palmarès mondial en nombre de millionnaires. Dans ces conditions, comment pouvez-vous encore nous faire croire que nous ne pouvons pas lutter efficacement contre la précarité qu'il n'est pas possible de garantir des conditions de vie dignes à l'ensemble de nos concitoyens ? L'État doit se mettre au service de nouveaux droits sociaux, de nouveaux droits environnementaux, plutôt que de les assécher par une déresponsabilisation générale en distribuant exonérations de cotisations et niches fiscales à tout-va, sans percevoir l'embrasement inévitable. La responsabilisation, ce gouvernement n'a eu que ce mot à la bouche,

mais restait aveugle à de graves failles de sécurité pourtant très visibles. » Plutôt que de nourrir les rancoeurs et les égoïsmes, défendons une République des communs, solidaire, qui aide véritablement les jeunes, renforce les moyens dans les écoles, investit dans les hôpitaux et donne des garanties aux élus locaux nous souhaitons lutter contre la fuite de capitaux, ce qui implique de ne pas réduire les effectifs du ministère de l'action et des comptes publics, comme le Gouvernement l'a fait. Tant de gabegies insupportables ! La privatisation d'Aéroports de Paris, justifiée par la création d'un fonds inutile, en est une belle illustration. La stratégie du tâtonnement du Gouvernement révèle son absence de vision. Sa politique austéritaire est inefficace, tant pour réduire le déficit que pour soutenir l'action publique. L'État agit aujourd'hui

compte tenu de la distance qui les sépare de la Terre, que ces astres ont parfois disparu au moment où nous apercevons la lueur qu'ils diffusaient. Entre l'instant où le signal lumineux a été émis et celui où il est reçu, la situation a eu le temps de changer ainsi que nous observons une situation qui n'est déjà plus. Tel est, en quelque sorte, l'effet que produit le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes pour 2019 : il nous rappelle cette époque, pas si éloignée, mais qui nous paraît déjà lointaine, où la France connaissait la croissance, réduisait son déficit public et maîtrisait son endettement. Cette impression est d'autant plus forte que nous venons de voter, dans la nuit de dimanche, le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Le déficit atteint désormais deux chiffres, le taux d'endettement a bondi de plus de 20 points et la dépense publique a franchi la barre des 60 % du PIB. La situation dont ce projet de loi rend compte n'a donc plus grand-chose à voir avec le présent. Mais il faut savoir tourner la page de 2019 pour affronter 2020 plus sereinement. C'est pourquoi le groupe Les Indépendants a considéré, dès la première lecture, qu'il valait mieux voter le projet de loi de règlement pour 2019. Il ne s'agit pas de donner un blanc-seing au Gouvernement pour sa politique économique. Il s'agit seulement de reconnaître le sérieux de sa gestion budgétaire. Il s'agit surtout de nous focaliser sur l'avenir, plutôt que de nous quereller sur le passé. Voter un texte budgétaire n'oblige pas à se satisfaire de la situation de nos finances publiques- je crois que la majorité des groupes sénatoriaux, en tout cas les groupes de la majorité sénatoriale, me rejoindront sur ce point. Ainsi, nous avons voté, il y a deux jours, le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, alors même qu'il sanctionne pour le pays une situation budgétaire catastrophique. Même si la situation budgétaire de 2019 nous paraît, avec le recul, enviable, je souhaite rappeler que la sonnette d'alarme avait déjà été tirée à plusieurs reprises. Bien sûr, le Gouvernement n'est pas seul responsable : la responsabilité est collective et partagée, puisque, depuis plus de dix ans, nous manquons de courage.

des précisions et nuances que je viens d'indiquer, nous considérons qu'il est important de reconnaître la bonne exécution de la loi de finances pour 2019. Mes chers collègues, les années qui sont devant nous s'annoncent difficiles.

l'échec de la commission mixte paritaire était prévisible, compte tenu des différences d'appréciation entre les assemblées, mais surtout de la superposition de ces textes et de ces débats.

Si nous nous penchons sur les comptes de 2019, que constatons-nous ? Oui, comme l'a souligné notre rapporteur général, le déficit était encore élevé, tutoyant la limite des 3 %, et la dette frôlait les 100 %, malgré des conditions économiques plutôt favorables en termes de croissance et des taux d'intérêt extrêmement bas, en contradiction avec la trajectoire des finances publiques sur le quinquennat. Tout cela est vrai, et nous en connaissons les raisons, à commencer par notre incapacité- j'utilise sciemment le nous collectif - à baisser durablement la dépense publique.

Depuis 2017, dans une période économiquement plutôt favorable où les recettes ont été systématiquement supérieures aux prévisions, et les intérêts de la dette inférieurs, c'est bien du côté des dépenses publiques que le bât blesse. En la matière, en dépit d'un certain nombre de réformes de compétitivité engagées, la situation n'a pas suffisamment évolué. Ainsi, l'année dernière, les dépenses ont encore augmenté de plus de 6 milliards le déficit structurel ne s'est pas réduit, comme l'a fait observer la Commission européenne. En conséquence, l'endettement de notre pays n'a pas été réduit au cours de cette période : il a continué son irrésistible progression, qui ne laisse pas d'inquiéter. Certes, les comptes publics ont été aggravés notamment par la crise des « gilets jaunes », qui a conduit le Gouvernement à ajouter en urgence des dépenses qui n'étaient pas prévues initialement. Le Sénat a d'ailleurs voté ces mesures pour mettre fin à la crise sociale dans le pays- souvenons-nous-en.

reconnaître également, comme nous l'avons tous fait, les efforts du Gouvernement en matière de sincérisation des comptes publics, de transparence et de bonne exécution des crédits ; je pense à l'absence de décret d'avance et à la mise en réserve de crédits réduite. Il faut le reconnaître dans un projet de loi qui traduit l'exécution du budget : souvenons-nous des périodes antérieures, pas si lointaines, où les budgets qui nous étaient présentés en loi de finances initiale n'étaient pas totalement sincères et réalistes. Toujours est-il que les difficultés demeurent- on le constate aujourd'hui, où nous subissons une crise hors du commun. entrés dans cette crise avec des comptes publics encore dégradés et une situation budgétaire plus dégradée que celle de la plupart de nos voisins européens, nous nous retrouvons dans une situation délicate, au moment où tous les États doivent emprunter massivement pour soutenir l'économie et faire face à des dépenses contraintes. Comme en première lecture, le groupe Union Centriste s'abstiendra sur ce texte, compte tenu de l'appréciation équilibrée qu'il porte sur l'exécution du budget 2019 et en considérant que le débat doit désormais porter sur les modalités de la nécessaire relance de l'activité

le souligner. Toutefois, si le groupe socialiste et républicain n'avait pas adopté la loi de finances initiale pour 2019, ce n'était pas pour les raisons développées par la majorité sénatoriale

Tous les indicateurs démontrent que l'appauvrissement de certains de nos concitoyens s'est aggravé, au bénéfice des plus aisés. Dès lors, nous continuerons de réitérer nos propositions pour une taxation rénovée de la fortune et du capital, dont vous ne voulez pas entendre parler. En matière de dépenses, nous considérons que les choix opérés en 2019 ont été insuffisants, notamment dans les domaines de la santé et de l'hôpital et de la lutte pour relever le défi environnemental, mais aussi de la solidarité à l'égard des territoires pour réduire les fractures sociales territoriales. Au titre des dépenses utiles, nous rappelons que la transition énergétique est un formidable levier de création d'emplois non délocalisables et bons pour notre planète et notre santé. Tout le monde le reconnaît, mais nous attendons les actes concrets

L'éducation, tout comme l'enseignement supérieur et la recherche, devra être dotée correctement pour préparer l'avenir du pays ; nous attendons le plan de relance à cet égard. Enfin, la culture, le tourisme et le sport, vecteurs d'emplois et de cohésion sociale, ne doivent pas être négligés,

Je vais vous le démontrer. Je suis allé rechercher ce qui figurait dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017, et j'y ai trouvé deux petits passages que je vous cite. Sous un chapitre intitulé « La préparation de l'avenir », on lisait : « Ne pas réduire nos dépenses courantes et notre dette serait irresponsable pour les générations à venir. » Voilà ! Tout à fait d'accord ! Un peu plus bas, on lisait : « Un plan d'économies sera mis en oeuvre au cours du quinquennat. Il permettra, à l'échéance du quinquennat, en 2022, d'économiser 60 milliards d'euros par an

Vous avez renoncé, alors que notre économie était en haut de cycle ; il y avait donc, peut-être, quelques marges de manoeuvre à exploiter. Malheureusement, cela fait deux ans que notre déficit structurel se situe à 2,2 %. Aucun effort n'a donc été fait, et nous n'avons même pas respecté la loi de programmation des finances publiques.

notamment à la faiblesse des taux d'intérêt, ce qui vous permettait,, en termes d'affichage, de dire que les choses s'amélioraient. Mais, à regarder strictement le budget de l'État, je suis désolé de vous dire qu'il n'y avait eu aucune amélioration jusqu'en 2019, et que les choses s'étaient même sérieusement dégradées.

Et, malheureusement, chacun l'a dit, avec la crise du covid, les choses ne peuvent plus s'améliorer. Tout ce que nous pouvons espérer maintenant, c'est de limiter les dégâts. Notre taux d'endettement avait atteint 98

l'article 6. Je vais mettre aux voix l'article 7. Je rappelle que, si cet article n'était pas adopté, il n'y aurait plus lieu de voter sur l'ensemble du projet de loi, dans la mesure où tous les articles qui le composent auraient été supprimés. Or, en application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit sur l'ensemble du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2019. En conséquence, l'article 7 va être mis aux voix par scrutin public.

la parole ? ... Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

sept articles du projet de loi ayant été successivement rejetés par le Sénat, je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire, puisqu'il n'y a plus de texte. En conséquence, le projet de loi de règlement

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 2 juillet dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun sur la proposition de loi permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19. Cet accord, qui est le fruit d'échanges constructifs avec notre collègue député Christophe Blanchet, auteur et rapporteur du texte pour l'Assemblée nationale, devrait nous conduire à adopter définitivement cette proposition de loi, qui vise à organiser les manifestations de générosité des Français en direction des personnels soignants mobilisés au plus fort de la crise sanitaire. Je tiens cependant à rappeler, s'agissant de la forme, que ce texte a été inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée par le précédent gouvernement, qui a décidé d'engager la procédure accélérée pour son examen, alors que le Parlement

cette proposition de loi, qui répond certes à une intention généreuse, ne correspond pas- nous en sommes tous conscients -aux attentes et aux revendications des personnels soignants ; le Ségur de la santé a d'ailleurs parallèlement été négocié à cette fin. Par ailleurs, il me semble que les moyens par lesquels nos concitoyens peuvent se montrer solidaires, notamment en donnant du temps ou de l'argent, sont suffisamment nombreux dans notre pays, et qu'il n'est pas urgent de légiférer à ce sujet. Au demeurant, si les personnels soignants méritent très certainement notre reconnaissance, ils ne sont évidemment pas les seuls à avoir pris des risques en travaillant pendant la période de crise sanitaire. À l'inverse, certains de nos concitoyens auraient aimé pouvoir continuer à travailler, mais se sont trouvés privés de cette possibilité. Enfin, je rappelle que nous avions été saisis d'un texte inabouti, dont tous les paramètres devaient être précisés ultérieurement, par voie réglementaire. On nous demandait donc de voter un principe, certes intéressant, sans avoir la moindre information sur les modalités de mise en oeuvre envisagées. Cependant, soucieuse de ne pas rejeter purement et simplement un texte favorable aux personnels soignants, la commission des affaires sociales, suivie par le Sénat, a réécrit ledit texte afin de le rendre plus opérationnel. Le dispositif de don de jours de repos imaginé par les députés, qui revenait dans bien des cas à demander aux employeurs, notamment publics, d'être généreux à la place de leurs salariés ou de leurs agents, a ainsi été remplacé par un mécanisme de don concret d'une partie de la rémunération du salarié correspondant à une ou plusieurs journées de travail. Le texte de la commission mixte paritaire qu'il vous est aujourd'hui proposé de voter est un compromis entre ces deux positions. Il conserve les apports du Sénat tout en rétablissant la possibilité, chère à l'Assemblée nationale, mais qui nous était apparue complexe, de monétiser des jours de repos. Cette possibilité demeure soumise- et cela me semble essentiel -à l'accord de l'employeur. Cette précision permettra de ne pas mettre en difficulté les employeurs, notamment publics, qui n'auraient pas les moyens de financer la générosité souhaitée par leurs salariés ou leurs agents. En outre, le texte de la commission mixte paritaire permet à toute personne physique ou morale d'abonder directement ce fonds par un don financier, ce que prévoyaient aussi bien le texte du Sénat que celui de l'Assemblée nationale. C'est là, en définitive, la manière la plus simple de contribuer à ce fonds, si bien qu'il s'agit peut-être de la disposition la plus prometteuse de la proposition de loi. Le texte adopté en commission mixte paritaire reprend par ailleurs l'essentiel des apports du Sénat visant à encadrer le dispositif. ainsi bénéficier des chèques-vacances les personnels des établissements et services sanitaires, médico-sociaux et d'aide à domicile ayant travaillé pendant la période du 12 mars au 10 mai 2020, qui correspond à la période de confinement de la population, et dont la rémunération est inférieure à trois fois le SMIC. Le principe, introduit par le Sénat, de la fixation d'une date limite pour faire un don dans le cadre de ce dispositif est également maintenu. Compte tenu de l'urgence dans laquelle le Gouvernement nous demandait de nous prononcer, nous avions fixé cette date au 31 août. La commission mixte paritaire a finalement retenu la date du 31 octobre prochain. De même, la date butoir pour la distribution des chèques-vacances, introduite par le Sénat, est conservée. Ainsi, les sommes versées à l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) qui n'auraient pas été distribuées sous forme de chèques-vacances au 31 décembre 2020 seront reversées au Trésor public. Nous avons par ailleurs accepté certaines modifications du texte adopté par le Sénat. Afin de mettre en oeuvre ce mécanisme de don le plus vite possible, le texte renvoie la détermination de ses modalités d'application à un décret simple au lieu d'un décret en Conseil d'État. Les modalités de répartition des chèques-vacances entre établissements seront également déterminées par décret, étant précisé qu'elles devront tenir compte des effectifs des établissements et services concernés. Malgré notre travail de précision,

avant le 31 mars 2021, sur les sommes qui auront été récoltées et sur la manière dont elles auront été réparties. Si ces sommes sont substantielles, tant mieux.

Madame la présidente, madame la rapporteure Frédérique Puissat, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureuse d'être parmi vous à l'occasion de la lecture des conclusions de la commission mixte permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19 est long, certes, mais il résume à mon sens très bien l'esprit et l'intention de ce texte. Je suis heureuse, d'abord, de voir consacrer une forme de solidarité essentielle, celle dont nous souhaitons témoigner envers nos soignants. Ils ont été en première ligne face au covid, et- nous le savons tous -, bien qu'ils l'aient parfois fait au péril de leur vie ou à l'épreuve de leur santé, jamais ils n'ont compté leurs heures ou économisé leur énergie. En tant qu'élue locale, j'ai eu l'occasion d'aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes particulièrement investis et de leur témoigner ma reconnaissance et celle de la Nation. Ils m'ont fait part de la difficulté à vivre ces moments douloureux qui les marquent à jamais. J'ai, ce soir, une pensée pour toutes celles et pour tous ceux qui ont été frappés par la maladie, et pour toutes celles et pour tous ceux qui ont perdu un proche. Naturellement, face à l'engagement sans faille du personnel soignant, nos concitoyens ont cherché à les remercier pour leur sacrifice et pour leur engagement. Après les applaudissements, certains ont donc souhaité aller plus loin et pouvoir donner des jours de congé aux personnels soignants. Cette proposition de loi vient justement consacrer une forme de solidarité nouvelle envers les soignants, salariés et non-salariés, du secteur public comme du secteur privé, y compris étudiants, afin qu'ils puissent eux aussi se reposer, profiter de leur famille, prendre des vacances et s'accorder des loisirs : retrouver, retrouver, en somme, un peu de légèreté et, surtout, prendre un peu de temps après le tsunami qu'a représenté le virus. Cette proposition de loi répond ainsi à une double attente, celle de nos concitoyens de créer de nouveaux mécanismes de solidarité, et celle des soignants de pouvoir en bénéficier. En ayant su entendre et traduire par la loi ces attentes fortes, le Parlement a une nouvelle fois illustré son rôle primordial de relais des préoccupations des Français et d'acteur essentiel de notre vie démocratique. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, je suis une élue locale : cela façonne ma pensée, ma méthode et aussi mon action. Je ne peux que saluer le choix qui a été fait par le Parlement de s'inspirer d'un mécanisme qui existait déjà et qui fonctionne celui du don de jours de repos, jusqu'alors réservé aux personnes ayant la charge d'un enfant gravement malade ou aux proches aidants. C'est là, je le crois, la clé de la réussite : s'inspirer de ce qui existe déjà et fonctionne pour le reproduire, l'élargir ou l'adapter. Nous pouvons saluer les mécanismes complémentaires et innovants que prévoit ce texte. Afin de permettre au plus grand nombre de déclencher un don de jours de repos, le Parlement a conçu plusieurs dispositifs

je l'ai dit, ce texte répond à une double attente. Pour être tout à fait précise, sans doute devrais-je dire qu'il répond en réalité à une attente supplémentaire celle de soutenir un secteur lui aussi très durement touché par la crise, le secteur du tourisme. Le don de jours de congé étant adossé aux chèques-vacances, c'est bien un soutien au tourisme qui est proposé. Ainsi, c'est bien d'une pierre deux coups que cette proposition de loi tend à apporter des réponses à la crise sanitaire et économique que nous traversons. Naturellement, cette proposition de loi n'a nullement vocation à se substituer aux politiques publiques, ni dans le domaine de la santé et du médico-social ni dans celui du tourisme. Ce sont bien les politiques publiques qui doivent dès aujourd'hui répondre aux difficultés structurelles de ces deux secteurs. Personne, d'ailleurs- je le crois -, ne dirait l'inverse : l'accord majoritaire des syndicats avec le Gouvernement sur le Ségur de la santé en est le marqueur le plus clair. À l'issue de la crise, c'est un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières qui est déployé. Nous parlons ici de 8,1 milliards d'euros qui bénéficieront à 1,8 million de professionnels. De même, pour ce qui concerne le tourisme, le lancement du plan de soutien interministériel au tourisme annoncé le 14 mai dernier par le Premier ministre est une réponse d'une ampleur inédite apportée par le Gouvernement à ce secteur particulièrement frappé par la crise, ce plan étant crédité de 18 La Nation, par l'hommage aux soignants voulu par le Président de la République le 14 juillet, a pu symboliquement leur témoigner sa reconnaissance. Il y avait là une première étape, essentielle à la reconnaissance de ce que nous leur devons collectivement. Les mesures prises par le Gouvernement pour répondre aux difficultés structurelles et à l'urgence représentent une seconde étape. Je souhaite saluer le travail de Mme la rapporteure, Frédérique Puissat, et de l'ensemble des groupes parlementaires et des sénateurs sur ce texte, qui s'inscrit dans une logique d'écoute des demandes de nos concitoyens et de solidarité nationale envers nos soignants au bénéfice des acteurs du tourisme.

En effet, au cours des derniers mois, au plus fort de la crise, les Français n'ont eu de cesse que d'inventer de nouvelles générosités pour apporter un soutien moral aux soignants sous pression face à l'épidémie de la covid-19. Applaudissements, livraisons de repas chauds dans les services les plus tendus des hôpitaux ... : nous savons tous que ces manifestations sont allées droit au coeur des soignants. Personnels des secteurs sanitaire et médico-social, personnels des hôpitaux, des établissements pour personnes âgées ou des services à domicile et personnels non salariés, qu'ils soient soignants ou non, ont tous multiplié les heures de travail sans prendre de repos, faute de personnel disponible pour les relever, ou, simplement, par esprit de dévouement professionnel. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons également du fait que le Gouvernement ait engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi, puisqu'il s'agissait de ne pas déconnecter le mécanisme ainsi proposé de la situation de crise. Bien évidemment, j'y insiste, notre travail de législateur n'est pas de faire des lois d'émotion. Pour autant, lorsqu'une pandémie d'une ampleur sans précédent nous frappe, nous ne pouvons rester insensibles aux besoins affichés par nos concitoyens.

C'est donc dans un double objectif que l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi de Christophe Blanchet : faire un geste original envers le personnel soignant en offrant un ou plusieurs jours de repos sous forme de chèques-vacances et permettre aux Français qui le souhaitent de faire un geste de solidarité- c'est peut-être là l'essentiel. La proposition de loi comportait initialement un système de don de jours de repos qui n'a pas satisfait la majorité sénatoriale, sous prétexte qu'il paraissait complexe à mettre en oeuvre. Dans le texte qui résulte des travaux du Sénat, il n'était donc plus question de don de jours de repos, mais de don d'une partie de la rémunération du salarié correspondant à un ou plusieurs jours de travail : en d'autres termes, une retenue sur salaire.

Il est en outre précisé qu'un accord d'entreprise pourra prévoir un abondement de la part de l'employeur. Je ne reviendrai pas sur toutes les précisions qui ont été apportées au cours de la navette parlementaire ou par la commission mixte paritaire, mais je tiens à rappeler que nous avons délimité dans le temps la période durant laquelle les personnels devront avoir travaillé pour bénéficier des chèques-vacances-

réintroduit le don de jours de repos, offrant ainsi deux possibilités plutôt qu'une au salarié et à l'employeur- nous nous réjouissons que cette alternative ait finalement été intégrée : elle contribue à l'ouverture du dialogue social dans l'entreprise. Bien entendu, cette proposition de loi n'est en aucun cas destinée à se substituer aux politiques publiques qui visent à apporter une réponse pérenne aux difficultés structurelles des secteurs de la santé et du médico-social. Est-il nécessaire de rappeler les chantiers engagés avant la crise sanitaire le plan Ma santé 2022 ? Est-il nécessaire de rappeler, une semaine après la signature des accords sur les salaires avec les syndicats, les propositions dévoilées hier matin par le Gouvernement, à l'occasion de la clôture du Ségur de la santé, pour améliorer le fonctionnement et l'organisation du système de soins ? et l'organisation du système de soins ? Près de 2 millions de personnels sont concernés par les revalorisations salariales, dont plus de 1,5 million de professionnels non médicaux dans les hôpitaux publics, les Ehpad et les structures privées à but non lucratif. Concrètement, la revalorisation « socle » prévoit une hausse de 183 euros nets mensuels pour les professionnels de l'hôpital et des Ehpad publics, hors médecins. L'accord prévoit également une refonte des grilles salariales de la fonction publique qui portera la revalorisation à plus de 200 euros nets mensuels. Une évolution plus dynamique des carrières est ainsi prévue. Le Premier ministre s'est également engagé sur le recrutement de 15 000 postes, ce qui n'est pas anodin. L'accord signé avec les médecins hospitaliers porte sur une enveloppe globale de 450 millions d'euros. Cette enveloppe servira essentiellement à doubler l'indemnité de « service public exclusif » versée aux praticiens qui s'engagent à ne travailler que dans les hôpitaux publics. est aujourd'hui de 490 euros bruts par mois. Elle passera à 1 010 euros pour tous les praticiens éligibles, en deux temps. Quant aux internes, ils vont bénéficier d'une enveloppe de 124 millions d'euros ainsi que de mesures visant à assurer un meilleur respect de leur temps de travail. Cette enveloppe, qui permettra d'améliorer les indemnités versées aux jeunes praticiens, répond à une revendication de longue date des futurs médecins. Mes chers collègues, les trente-trois grandes orientations du Ségur de la santé, présentées hier, trouveront bientôt une traduction réglementaire et législative, dans le projet de loi de Si de nombreux défis doivent encore être relevés, le cap ambitieux qui a été choisi doit être accompagné ! Notre groupe sera à la hauteur du moment. Vous l'aurez compris : cette proposition de loi ne saurait en rien se substituer à la réforme profonde du système de santé engagée par le Gouvernement. Elle n'est qu'un « plus

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, alors que le Gouvernement vient de dévoiler le second volet des mesures du Ségur de la santé, nous considérons que les annonces ne sont pas à la hauteur des attentes. Le Gouvernement a annoncé 2 milliards d'euros sur cinq ans pour la transformation, la rénovation et l'équipement des établissements médico-sociaux, c'est une première étape nécessaire, mais insuffisante pour rattraper le retard accumulé. retard accumulé. Le Premier ministre a promis une augmentation de salaire des personnels des hôpitaux et des Ehpad publics de l'ordre de 183 euros nets mensuels. Nous sommes bien loin du rattrapage et de la reconnaissance attendus, et en deçà des 300 euros réclamés par tous les syndicats pour que la France ne soit plus la mauvaise élève de l'OCDE. Cette augmentation ne sera d'ailleurs pas immédiate puisqu'elle devra encore être votée lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. En attendant, le ministre de la santé a annoncé la création de 15 000 postes alors que les syndicats des hospitaliers chiffrent les besoins à 100 000 postes. C'est un premier pas, mais nous sommes encore loin de la reconnaissance des personnels des secteurs sanitaire et médico-social pour leur engagement au quotidien, particulièrement durant la crise du covid-19. Mais nous sommes également encore loin du choc d'attractivité dont a besoin l'hôpital. Comme je l'avais indiqué en première lecture, les personnels manquent non pas de congés, mais d'effectifs pour pouvoir poser des jours ! Les personnels ne demandent pas la charité, ils souhaitent simplement pouvoir se reposer en utilisant leurs propres jours de congé. Pour y parvenir, il faut avoir des collègues et pas des postes vacants. La commission mixte paritaire a trouvé un accord sur la proposition de loi en retenant la rédaction de la droite sénatoriale, pourtant très différente de celle de la droite de l'Assemblée nationale. Désormais, nous ne parlons pas d'un texte qui permet les dons de jours de repos, mais d'un texte qui permet les dons de journées de travail. La différence n'est pas neutre, surtout quand on examine dans moins d'une heure un texte sur la dette sociale et la création d'une branche relative à la perte d'autonomie. Le don de journées de travail existe déjà puisque tous les travailleurs, à l'occasion de la journée de solidarité, ont le choix entre donner à leur employeur une journée de travail ou donner une partie de leur salaire au profit du financement des retraités. Disons-le tout de suite, notre groupe s'était opposé à la création de la journée de solidarité. Nous nous opposerons à d'éventuelles tentatives d'ajouter des mardis ou des mercredis de Pentecôte En tout état de cause, le fait pour un salarié de pouvoir donner une partie de son salaire ou des jours de repos est une fausse solidarité. C'est une aide entre travailleurs et cela s'appelle le syndicalisme. Si cela peut sembler bien curieux pour la droite sénatoriale, nous sommes, pour notre part, habitués à soutenir les caisses de grève des salariés en lutte pour leurs droits. La véritable solidarité, c'est lorsque des personnes aux intérêts divergents s'unissent. En ce qui concerne les personnels médicaux ou paramédicaux, une véritable solidarité

au 31 décembre 2020 dans les caisses des finances publiques où il pourra véritablement servir l'intérêt général. Par conséquent, notre groupe votera contre cette proposition de loi. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « on ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout écrivait l'abbé Pierre, dont la sagesse n'avait d'égale que l'humilité. La proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui pour approbation est une belle illustration de cette phrase. cette phrase. Ce texte modeste, mais utile, vise à proposer à chaque salarié volontaire d'offrir des jours de congé sous la forme de chèques-vacances aux soignants et aux personnels médico-sociaux qui ont démontré leur engagement au service de la santé des Français durant la période de confinement. Si ces dispositions ne vont pas révolutionner la vie des soignants, peut-être permettront-elles d'améliorer à la marge leur pouvoir d'achat. Il s'agit d'un geste de solidarité individuelle, qui ne saurait en aucun cas se substituer à la solidarité nationale ni aux mesures gouvernementales. Ces dispositions proviennent d'une initiative citoyenne qu'il convient de rappeler. Le 20 mars dernier, le groupe Pasteur Mutualité a lancé la campagne « Je donne mes RTT » sur les réseaux sociaux, s'inspirant du dispositif existant pour les proches aidants. La proposition de loi vise à traduire dans notre législation une pratique inaugurée par un certain nombre d'accords d'entreprises depuis le début de l'épidémie. Ces initiatives sont de deux ordres : d'une part, une solidarité interne, permettant aux salariés de s'entraider au sein d'une même entreprise pour réduire les conséquences de l'activité partielle ; d'autre part, une solidarité externe qui s'exprime par le don de jours de repos monétisés puis reversés à des associations de soutien aux soignants. Or le cadre législatif actuel dû, notamment, à l'initiative de deux députés du Nord, Paul Christophe et Guy Bricout, se limite au don de jours de congé monétisés aux parents d'un enfant gravement malade et à un proche aidant. il s'agit d'accompagner le volontarisme d'un certain nombre d'entreprises en adaptant notre législation, de façon provisoire, à la situation d'exception que nous avons traversée ces derniers mois. Si la loi n'a pas vocation à être le réceptacle de mesures provisoires, il me semble qu'elle ne doit pas faire obstacle aux initiatives citoyennes. Dans un contexte de fortes tensions économiques, il serait inconvenant de décourager les élans de solidarité individuelle. C'est pourquoi notre groupe se félicite du succès de la commission mixte paritaire, réunie en urgence le 4 juillet dernier. Nous saluons le travail réalisé pour préserver les avancées apportées par le Sénat tout en maintenant dans la loi le dispositif de dons de jours de congé proposé initialement par l'auteur de ce texte, le député Christophe Blanchet. Dans une démarche constructive, la commission des affaires sociales du Sénat a proposé, en première lecture, de réécrire l'article 1 pour remplacer le don de jours de congé par le versement d'une partie de la rémunération du salarié correspondant à une ou à plusieurs journées de travail. Le dispositif final a préservé l'esprit initial de la proposition de loi en conjuguant les deux possibilités de don, sous forme de jours de congé et sous forme d'un montant correspondant à la rémunération perçue au titre d'une ou de plusieurs journées de travail. Le Sénat a également proposé de borner le dispositif dans le temps, posant l'échéance du 31 août de façon à circonscrire les dons au plus près de la période de confinement. La commission mixte paritaire a préservé ce bornage temporel tout en étendant l'échéance de versement des dons au 31 octobre 2020, ce qui me semble être un bon compromis pour laisser le temps aux salariés de s'approprier le dispositif. Enfin, il a été convenu de renvoyer les modalités de la répartition des dons à un décret simple afin d'accélérer l'application de la loi. Les principales avancées du Sénat sont maintenues tout en préservant l'esprit du texte initial. Nous voterons donc les conclusions de la commission mixte paritaire.

Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19. Je m'associe à l'hommage que vous leur avez rendu, chacun se reconnaîtra dans les mots que vous avez prononcés. La commission mixte paritaire, qui s'est tenue le 2 juillet dernier, a abouti à un accord. Je m'en réjouis. Je souligne que celle-ci s'est réunie très rapidement, à peine plus d'un mois après le dépôt du texte à l'Assemblée nationale.

en vacances- certains en ont vraiment besoin -et cette proposition de loi est clairement à contretemps. L'échéance initialement proposée du 31 août 2020 était certainement trop brève pour permettre au dispositif d'être efficace en suscitant un nombre de dons suffisant.

plus vite possible. Nous arrivons là aux limites de l'exercice. L'élaboration d'une loi par le Parlement nécessite du temps. Nos procédures ne permettent pas de réagir aussi rapidement que nécessaire.

Sinon, je crains que cette proposition de loi ne soit d'ores et déjà mort-née. Rappelons-nous les mots de Montesquieu : « Il ne faut point faire par les lois ce que l'on peut faire par les moeurs. Or des initiatives locales ne nous ont pas attendus pour saluer les héros de cette crise. Avec la campagne intitulée « le repos des héros », un certain nombre d'organismes de tourisme se sont mobilisés, sous l'impulsion des collectivités,

la ministre, ont ouvert ces bons-vacances à d'autres corps de métier particulièrement exposés, comme les hôtes de caisse, ce qui fait défaut à cette proposition de loi qui n'intervient que pour un seul Tout comme le dispositif qui nous est soumis aujourd'hui, cette initiative vise à soutenir les professionnels du tourisme dans la relance de leur activité, tout en remerciant nos héros qui ont besoin de se ressourcer. Enfin, il est à noter que les tirages au sort se sont tenus dès le début du mois de juin. Des centaines de soignants ont donc certainement déjà profité de ces séjours. La seule limite réside dans ce système injuste de tirage au sort. Un système plus Un système plus universel aurait pu être mis en oeuvre en partenariat avec les pouvoirs publics, sans forcément passer par une loi. Sur le fond, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire combine les dispositifs adoptés par l'Assemblée nationale Un salarié pourra donc soit donner une partie de son salaire, notamment s'il ne dispose pas de jours de RTT, soit donner les jours de repos qu'il a pu accumuler sur un compte épargne-temps, par exemple, en accord avec son employeur.

L'acquisition de ces chèques-vacances est exonérée de l'impôt sur le revenu, ce qui est une très bonne chose. Enfin, le Gouvernement devra remettre un rapport au Parlement d'ici au 31 mars prochain afin de s'assurer de l'application réelle du dispositif et de retracer la distribution des chèques-vacances

avec un niveau d'engagements financiers inédit. À ce stade, le Ségur mobilisera plus de 28 milliards d'euros, soit 9,1 milliards pour le fonctionnement et 19 milliards pour l'investissement, dont 13 milliards d'euros de reprise de la dette des hôpitaux.

Hier, le ministre présentait les conclusions, très attendues de ce Ségur, davantage consacré aux réformes structurelles. Nous resterons vigilants quant à l'application de ce dispositif dans les territoires. Les hôpitaux, et plus largement les établissements, ne sont pas les seuls acteurs de l'offre de soins. soins. Je salue la volonté du ministre d'associer davantage les élus, la médecine de ville et l'ensemble des parties prenantes à cette refonte fondamentale de notre système de santé. Enfin, le groupe Union Centriste a pris part à cette concertation en transmettant au Premier ministre ses réflexions sur deux sujets centraux, la gouvernance de notre système de santé et la place de nos aînés, qui posent assurément les jalons d'une politique sanitaire plus décentralisée et plus humaniste que nous appelons de nos voeux. Je terminerai en reprenant les mots de ma collègue Jocelyne Guidez : « Il ne serait pas envisageable un seul instant de voter contre cette mesure de solidarité ». Aussi, le groupe Union Centriste votera cette proposition de loi en espérant que cette belle intention soit réellement utile

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes de nouveau invités ce soir à discuter de la proposition de loi visant à permettre d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19. Je ferai tout d'abord quelques remarques sur les modifications apportées en commission mixte paritaire. Premièrement, la possibilité de monétiser des jours de repos non pris, supprimée au Sénat, a été réintroduite et vient se superposer au mécanisme de renonciation à la rémunération d'un ou de plusieurs jours ouvrés. Nous le jugeons regrettable, car le rapport de notre collègue rapporteur Frédérique Puissat était pourtant on ne peut plus clair à ce sujet : quand bien même le mécanisme de monétisation des jours de congé serait précisé par la proposition de loi, ce qui n'est pas le cas,

De la même manière, la modification opérée quant aux modalités de répartition des sommes réunies reste insatisfaisante en l'état. D'une part, il est difficile de juger en quoi il serait plus pertinent que la répartition s'opère selon les effectifs plutôt que selon la masse salariale. D'autre part, le renvoi à des décrets signe l'incapacité à construire un cadre légal à la hauteur de l'objectif initial. Deuxièmement, les membres de la commission mixte paritaire sont tombés d'accord pour exonérer l'acquisition de chèques-vacances de l'impôt sur le revenu. Il est cependant curieux de constater que cette exonération ne concerne que l'acquisition des chèques-vacances et non le don qui, lui, reste intégralement soumis à l'impôt.

la raison pour laquelle nous jugeons étrange, par ailleurs, de prévoir un reversement au Trésor public des sommes non distribuées. Fallait-il, dans ce gloubi-boulga, que le Trésor public y trouve son compte ?

Sur la forme, et dans un contexte de précipitation de la part du Gouvernement pour faire adopter cette proposition de loi, celle-ci demeure dans sa rédaction finale incomplète, floue, complexe à mettre en oeuvre et très probablement promise à l'insuccès. Quant au fond, les principales sources de trouble sont toujours bien présentes. Tout d'abord, comme cela a été rappelé, les soignants sont les seuls concernés par cet élan de générosité que vous prétendez faciliter. Ils font part, eux-mêmes, de ce sentiment de gêne, car des travailleurs et travailleuses de beaucoup d'autres secteurs- caissiers, livreurs, ouvriers, agents du service public -ont continué de travailler et ont affronté le risque de la contamination, parfois sans protection ; certains ont même été contaminés. Ensuite, cette proposition de loi suscite le doute au regard de la période actuelle marquée par une paupérisation grandissante d'une grande partie des Français. Le phénomène risque malheureusement de s'accroître à la rentrée. Vous habillez de valeurs de solidarité et de générosité une logique consistant à déshabiller Pierre pour habiller Paul, puisque vous demandez aux salariés de payer des chèques-vacances aux soignants.

le président, madame la ministre, chers collègues, moins de deux mois après l'engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement, nous devons aujourd'hui nous prononcer sur l'accord trouvé, en un temps record, par les députés et les sénateurs réunis en commission mixte paritaire. De par son contenu, cette proposition de loi nécessitait en effet une adoption rapide : étant en lien direct avec la crise sanitaire, repousser sa mise en oeuvre reviendrait à lui ôter toute forme d'utilité, utilité dont certains doutent déjà depuis le début de nos travaux Dès lors qu'elle recevait le soutien du Gouvernement, une mise en application rapide devenait possible. Grâce au travail constructif de nos deux assemblées, c'est devenu réel. Je tiens ainsi à saluer le travail de notre rapporteur, qui a permis d'aboutir à un compromis avec les députés, dans une temporalité particulièrement contrainte. Cette question de temporalité est souvent revenue lors de nos débats et de nos échanges. Elle continue de préoccuper un certain nombre d'entre nous. Alors que les soignants réclament à cor et à cri une réforme en profondeur du système de santé, il nous est apparu presque anachronique d'examiner en urgence une proposition modeste ou de petite envergure. Néanmoins, il n'a pas semblé opportun aux membres de mon groupe de s'opposer à l'adoption d'une mesure qui relèvera, pour les donateurs, du volontariat et, pour les bénéficiaires, d'un coup de pouce et d'une marque de reconnaissance bienvenus. Nous resterons naturellement sur cette même ligne aujourd'hui, d'autant que- comme je l'ai souligné lors de la discussion générale en première lecture -cette mesure permettra aussi de soutenir l'économie locale et le secteur du tourisme, qui en ont grandement besoin. Pour entrer plus en détail dans le coeur de la proposition qui nous est présentée aujourd'hui, nous nous réjouissons que, pour l'essentiel, les modifications du Sénat aient été conservées. Le dispositif prévoit ainsi, pour les salariés qui le souhaitent, le don d'une partie de leur rémunération, avec un abondement possible de l'employeur, et pour les non-salariés un don financier direct à l'ANCV, qui sera chargée de transformer ces sommes en chèques-vacances. Tous les personnels du secteur sanitaire et médico-social pourront en bénéficier, à condition qu'ils aient travaillé pendant la période de confinement et que leur rémunération ne dépasse pas trois SMIC. La date limite pour les dons est fixée au 31 octobre et la date limite pour la distribution des chèques-vacances est fixée au 31 décembre. Un rapport viendra, en mars 2021, détailler les sommes versées et la répartition des montants distribués. Cela nous permettra de vérifier si la loi a bien rempli son objectif. S'agissant d'une mesure qui n'a pas remporté une complète adhésion sur ces travées, et compte tenu de la complexité du dispositif et des contraintes qui pèseront sur les entreprises, il est indispensable qu'un bilan en soit soit tiré. Nous saluons enfin l'ajout en commission mixte paritaire de l'exonération d'impôt sur le revenu pour l'acquisition de ces chèques-vacances. Il aurait été de mauvais ton de taxer les bénéficiaires sur des dons qui demeureront relativement modestes. Cela étant, si l'intention est louable- nous avons parlé à plusieurs reprises d'intention généreuse -, j'insiste sur le fait que les attentes des secteurs médical et médico-social sont immenses et légitimes, après des décennies de renoncement et de budgets contraints. Charge à nous et au Gouvernement de les respecter et de ne pas leur laisser croire qu'un chèque-vacance ou une médaille suffiront à rendre compte de la reconnaissance de la Nation. En effet, cette modeste mesure fait figure de goutte d'eau dans l'océan des besoins du monde médical. Le Ségur se termine. L'accord trouvé sur les revalorisations salariales est à saluer. Une grande marche a été franchie, qui permet de rattraper en partie le retard accumulé par rapport aux pays de l'OCDE sur la rémunération de nos soignants. Les récentes annonces du ministre de la santé font également espérer des réformes nécessaires dont le monde médical a tant besoin. Aussi, tout en votant cette proposition de loi et en saluant les premières avancées du Ségur, nous insistons sur le fait que les réformes doivent être mises en oeuvre au plus vite. vite. Je terminerai en rappelant que le succès de cette loi dépendra aussi de la promotion qui en sera faite par l'État. Pour que la mesure soit adoptée par le plus grand nombre, les pouvoirs publics doivent la faire connaître le plus largement et le et le plus rapidement possible compte tenu de la date butoir fixée au 31 octobre. Nous serons donc attentifs, madame la ministre, au travail déployé par vos services dans les prochaines semaines pour que les efforts mis en oeuvre par les parlementaires pour une application rapide de cette loi n'aient pas été vains. En cette période de vacances, que cette mesure permette à nos héros le repos tant mérité. Vous l'aurez compris, notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'examen de cette proposition de loi témoigne de l'élan de solidarité suscité par le dévouement des soignants ces derniers mois. Face aux difficultés qui se multipliaient, les personnels ont su faire front, et bien souvent s'oublier, pour gérer une crise sanitaire sans précédent. Entre autres manifestations de reconnaissance, l'idée d'offrir des jours de repos s'est exprimée, pour finalement se concrétiser dans le présent texte, qui permet également un mécanisme de conversion en chèques-vacances. Il faut souligner que cette proposition de loi inscrite en urgence, appuyée par le Gouvernement, a suscité une certaine incrédulité de la part des personnels concernés tant le décalage est important entre cet acte et leurs besoins réels, alors même que la plupart d'entre eux ne peuvent tout simplement pas prendre leurs jours de repos

Nous avons fait le choix de soutenir cette initiative. Il semble en effet difficile de se prononcer contre un texte solidaire. La proposition de loi permettra aux salariés français qui le souhaitent et le peuvent de témoigner leur reconnaissance, ce qui est important. Elle pourra également constituer, même si ce n'est pas son objectif principal et qu'il n'est pas certain qu'elle rencontre le succès escompté, un soutien au secteur du tourisme français, durement touché par la crise sanitaire. Le Sénat a donc choisi d'adopter une attitude constructive afin que le dispositif proposé puisse fonctionner sur le terrain, malgré une rédaction initiale approximative. La commission mixte paritaire, à laquelle j'ai participé, a conservé les principaux apports de notre Haute Assemblée. Il était notamment important de préciser que les bénéficiaires devront avoir travaillé pendant la période de confinement et de fixer une date limite pour faire un don dans le cadre de ce dispositif. Le Sénat a également prévu l'obligation de reverser au Trésor public les sommes versées à l'ANCV qui n'auraient pas été distribuées sous forme de chèques-vacances au 31 décembre 2020. Députés et sénateurs ont par ailleurs recherché une solution de compromis entre leurs positions respectives concernant le don de jours de repos non pris voté par l'Assemblée, à distinguer du don de rémunération privilégié par le Sénat. effet, pour notre rapporteur, dont je tiens à souligner la qualité du travail, réintroduire la perspective de dons de jours de repos est une source de complexité supplémentaire pour les entreprises une perte de sens, puisque le choix d'un salarié de renoncer à un jour de congé se traduira finalement par un versement de l'employeur. On aboutit alors à une sorte de prélèvement obligatoire pour l'employeur, ce qui s'éloigne de l'esprit de solidarité entre travailleurs qui motivait la démarche. Une rédaction de compromis a pu être trouvée permettant le don de jours de repos, mais en le conditionnant à un accord de l'employeur. Aussi les préoccupations des deux assemblées se trouvent-elles satisfaites. Il restera à vérifier si le dispositif atteint ses objectifs. Les préoccupations ont changé, certains salariés ont perdu des jours de congé ou rencontrent des difficultés financières. Le texte voté aujourd'hui sera-t-il utile dans ces conditions ? Malgré notre réticence à multiplier les rapports, conformément à une position constante du Sénat, nous avons décidé en commission mixte paritaire que le Gouvernement devrait remettre au Parlement un rapport retraçant l'ensemble des sommes allouées d'ici au 31 mars 2021. Notre groupe votera donc ce texte en espérant qu'il trouve à s'appliquer. Il faut s'attaquer maintenant aux vrais enjeux de notre politique de santé publique et éviter un simple saupoudrage de moyens financiers, comme le Gouvernement semble vouloir vouloir le faire à la suite du Ségur de la santé, même si des annonces plus systémiques ont été faites. Seules des réformes de fond pourront améliorer notre système de santé et répondre à l'investissement de nos soignants. La discussion

chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

du projet de loi relatif à la dette sociale et à l'autonomie (texte n° 661, 2019-2020) Il a été décidé que ces deux textes feraient l'objet d'une discussion générale commune.

Néanmoins, malgré des rapprochements et un souci commun, la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à s'accorder sur un texte identique. Je reviens donc devant vous en nouvelle lecture. Même si je comprends que l'examen des deux projets de loi sera raccourci, je souhaiterais dire quelques mots sur l'ambition pour l'autonomie que porte ce projet de loi. Cette ambition résulte en partie d'un amendement introduit par les parlementaires, qui visait à créer la cinquième branche de la sécurité sociale. J'ai suivi les débats qui se sont tenus dans cette chambre en première lecture et je comprends votre exigence visant à ce que cette disposition soit non pas seulement un effet d'annonce, mais bien la première pierre d'un grand projet. Cette création était attendue depuis longtemps. Je pourrais même dire qu'elle était évoquée depuis maintenant trois législatures. Vous reconnaîtrez que c'est là un tournant dans l'histoire de la sécurité sociale. Comme en 1945, quand il avait été décidé de créer une assurance sociale publique contre le risque de maladie ou d'accident du travail, le choix est aujourd'hui fait d'une nouvelle assurance publique contre ce qui est devenu un nouveau risque, auquel tous les Français peuvent être amenés Les chiffres sont sans appel, et je sais que sur ces travées vous les connaissez. Ils ont été récemment rappelés lors des travaux conduits l'année dernière par le sénateur Bernard Bonne et la sénatrice Michelle Meunier en 2040, près de 15 % des Français, soit 10,6 millions de personnes, auront 75 ans ou plus. C'est deux fois plus qu'aujourd'hui ! La création de cette branche permettra, d'abord, de donner toute la visibilité aux parlementaires, dès le projet sur son équilibre financier- je comprends que vous y serez vigilants. Pour autant, cette création n'est pas un point d'orgue, c'est bien le début du projet. Une mission vient d'être lancée, et elle rendra son rapport en septembre

les amendements qui ont permis de clarifier les modalités de consultation permettant d'élaborer ce rapport. Il est en effet essentiel que l'ensemble des acteurs soient associés soit trouvée une solution de consensus pour dégager au moins 1 milliard d'euros dès 2021, comme s'y est engagé le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, en première lecture. Je ne veux pas être trop longue, mais il me faut rappeler que ce texte est aussi une opération de bonne gestion, qui permet à la sécurité sociale de se refinancer sans s'exposer à un risque de taux ou de liquidité sur les marchés financiers. C'était même là son objectif principal. Avant de conclure, j'aimerais dire quelques mots sur la règle d'or, point sur lequel la commission mixte paritaire a échoué. Le Gouvernement a bien entendu la volonté d'encadrer les finances sociales, pour éviter que ne se reproduisent des déficits demain, la dette de nos enfants. Néanmoins, pour bien fonctionner, une règle d'or doit être crédible. Et pour assurer cette crédibilité, il faut un horizon d'équilibre. Aujourd'hui, et c'est la position que nous retenons, l'incertitude est trop forte et il est trop tôt. Le deuxième point d'achoppement, c'est la reprise de la dette hospitalière. Elle a été supprimée lors de l'examen dans cette chambre en première lecture, ce qui réduit de 13 milliards d'euros la marge d'investissement qui a été annoncée dans le cadre du Ségur En réalité, le déficit de l'assurance maladie et celui de nos hôpitaux sont liés- les économies de l'une ne peuvent se transformer en déficits des autres. C'est aussi cela que la reprise de cette dette traduit aujourd'hui. Enfin, le troisième point qui sera certainement abordé lors de la discussion générale concerne l'isolement de la « dette covid ». Le ministre l'avait dit lors de sa présentation, le traitement de cette dette est une question complexe, et encore largement débattue parmi les économistes, y compris les plus grands spécialistes des finances publiques. Le Premier ministre a indiqué lors de sa déclaration de politique générale vouloir en discuter avec les partenaires sociaux. Rien dans ce texte ne fait obstacle à l'isolement de la « dette covid », mais, en tout état de cause, il s'agit de répondre à l'urgence, ce qui a toujours guidé notre action. En conclusion, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaiterais vous faire part de mon état d'esprit, deux semaines après ma nomination en tant que ministre déléguée chargée de l'autonomie. Comme je le rappelais hier à l'Assemblée nationale, mon ambition, qui est celle du Gouvernement, est simple, mais elle se veut forte préserver le libre choix et surtout la dignité de nos compatriotes âgés. Vous en êtes conscients : la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et le soutien nous concernent toutes et tous, soit parce que nous connaissons un proche, un parent, affecté par cette perte d'autonomie, soit parce que, avançant en âge, nous nous posons des questions légitimes liées à cette dernière tranche de vie. Ce qui est en jeu est assurément humain, affectif et moral. Car c'est dans le sort qu'elle réserve, dans la place qu'elle donne, dans la considération qu'elle porte aux plus humbles, aux plus vulnérables, aux plus fragiles, que se mesure la valeur morale et humaine d'une société. Je suis convaincue que nous sommes en mesure de nous rassembler autour de cette belle ambition pour notre pays. Et je sais par avance que le Sénat, compte tenu de son lien charnel avec les territoires, de son expertise sur le sujet et surtout de l'exigence qui le caractérise, saura contribuer à enrichir ce beau projet par-delà les clivages partisans. Comptez donc sur moi, mesdames, messieurs les sénateurs, pour vous y associer à chaque étape. La parole

Pour ce qui concerne le volet relatif à l'autonomie, dont vous êtes chargée, les deux assemblées ont approuvé la création à venir d'une « cinquième branche Néanmoins, le Sénat souhaite qu'il y ait un véritable contenu derrière ce nom, en termes tant financiers que d'organisation. Nous attendons donc avec impatience les conclusions du rapport que le Gouvernement doit remettre au Parlement avant le 15 septembre. Nous notons également avec satisfaction que l'Assemblée nationale a retenu, en nouvelle lecture, les améliorations apportées par le Sénat afin de mieux encadrer le contenu du rapport et les consultations préalables à sa rédaction.

d'autre part, le report de la date limite d'extinction de la dette sociale au 31 décembre 2033, au lieu de 2024 comme cela était envisagé jusqu'à présent. Néanmoins, notre commission a dû constater qu'à côté de ces points d'accord, l'Assemblée nationale avait rétabli en nouvelle lecture sa version sur les deux points majeurs de divergence qui ont conduit à l'échec en commission mixte paritaire. Ainsi, à l'article 1 du projet de loi ordinaire, l'Assemblée nationale a réintroduit la prise en charge par la Cades d'une fraction de la dette des hôpitaux représentant un montant de 13 milliards d'euros. Or le Sénat s'était fermement, et presque unanimement, opposé à ce dispositif pour des raisons de fond que je rappelle brièvement : les hôpitaux ne sont pas la propriété de l'assurance maladie- on peut le regretter, mais c'est un autre sujet -, qui n'assure qui n'assure pas davantage la gestion de ces établissements. En outre, l'essentiel de la dette hospitalière provient d'investissements immobiliers lancés, notamment dans le cadre des plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012, sur l'initiative de l'État. Une telle situation créerait enfin, à nos yeux, un précédent dangereux qui pourrait être utilisé à l'avenir pour transférer n'importe quoi à la Cades, ce qui n'a pas échappé, semble-t-il, au Gouvernement, à en croire certains articles de presse. Il pourrait d'ailleurs être utile que le Conseil constitutionnel précise si un tel transfert de dette d'une personne autre que la sécurité sociale est bien compatible avec le principe constitutionnel d'équilibre financier de la sécurité sociale. Pour l'ensemble de ces raisons, la commission des affaires sociales et le Sénat dans son ensemble ont considéré qu'il appartenait à l'État d'assumer lui-même le coût de sa promesse, de l'automne dernier, de reprise d'un tiers de la dette des hôpitaux, que nous ne contestons pas,

dont nous étions prêts à débattre des modalités pratiques, l'Assemblée nationale ait suivi le Gouvernement. On peut en effet On peut en effet se demander si l'extinction de la dette sociale demeure réellement un objectif pour l'Assemblée nationale. Je ne mets pas en cause le Gouvernement. Il semble en effet paradoxal que le Premier ministre ait réaffirmé devant devant le Sénat, la semaine dernière, son souhait que les partenaires sociaux se saisissent, avec l'État, « des questions liées à l'équilibre de l'ensemble des régimes de protection sociale Si ce n'est pas une règle d'or, qu'est-ce donc ? Dans ces conditions, la commission des affaires sociales n'a pu que constater le caractère irréconciliable des divergences qui subsistent entre les deux assemblées et proposera donc au Sénat

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lors de la première lecture, j'avais eu l'occasion de présenter au nom de mon groupe une motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité constitutionnelle, car ce texte remet en cause l'autonomie de la sécurité sociale. Nous continuons à penser que ces deux projets de loi, organique et ordinaire, remettent en cause les fondements de la sécurité sociale. Cette étape supplémentaire vers une transformation de la « sécu » en filet de sécurité dépourvu de lien avec notre pacte social républicain est extrêmement grave. Derrière ces textes de loi, nous avons en réalité deux lois budgétaires à examiner. Tout d'abord, sur le transfert de 136 milliards d'euros à la Cades, nous contestons, avec la majorité du Sénat, le choix du Gouvernement de faire prendre en charge par cette caisse le financement d'un tiers de la dette des établissements de santé. Selon nous, la sécurité sociale n'a pas à assumer la dette des hôpitaux, qui provient principalement des investissements immobiliers. En effet, lorsque le précédent gouvernement avait annoncé une reprise de la dette, il n'avait pas mentionné que la dette reprise serait transférée à la Cades. La confusion que vous organisez, de plus en plus, entre le budget de l'État et celui de la sécurité sociale nous pose problème. Elle conduit en tout cas à un changement de l'organisation institutionnelle de notre pays, et cela mérite un débat plus poussé que celui que nous avons eu. La dette créée par la crise du covid-19 aurait dû appeler un débat budgétaire plus approfondi. De la même manière, je rappelle notre opposition à la tentative de la droite sénatoriale d'insérer une « règle d'or » dans les comptes sociaux pour les prochains projets de loi de financement de la sécurité sociale. Alors que nous avons pu constater l'importance de notre modèle de protection sociale lorsqu'il a fallu prendre en charge le chômage partiel des entreprises, mais également les faiblesses des hôpitaux auxquels on a imposé depuis vingt ans des budgets inférieurs aux dépenses, imposer une règle d'or reviendrait à sanctuariser l'austérité dans les dépenses sociales et donc à grignoter encore davantage sur les droits acquis.

Alors même que l'Union européenne a décidé, face à la crise, de laisser de côté les déficits des États, la droite sénatoriale veut transposer le modèle européen d'austérité dans notre sécurité sociale. Non seulement c'est complètement décalé, mais en outre, la droite sénatoriale devra assumer ce choix politique qui consiste à réduire les prestations de santé, les prestations familiales et les pensions de retraite et, plus généralement, l'ensemble des droits pour lesquels nos concitoyens ont cotisé. C'est elle qui sera responsable, demain, des lits supprimés, et des services fermés à cause de sa règle d'or ! Alors que le ralentissement économique entraîne une chute des rentrées de cotisations sociales, il y a urgence à dégager de nouvelles recettes plutôt que plutôt que de fermer le robinet des prestations sociales. Nous avons de nombreuses propositions de recettes, mais vous refusez d'ouvrir le débat sur l'efficacité des exonérations de cotisations sociales. Plutôt que de faire peser le remboursement des 136 milliards d'euros sur les assurés sociaux par la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), on aurait pu imaginer un financement de la perte d'autonomie par les entreprises, en particulier celles qui font des milliards d'euros de bénéfices sur le dos de nos aînés. Le deuxième volet de la réforme est une véritable opération de communication. Alors que la crise sanitaire a démontré l'importance d'une intervention publique pour les personnes en perte d'autonomie dans les Ehpad ou à domicile, vous proposez une cinquième branche de la sécurité sociale sous-financée, qui ne permettra pas de réduire le reste à charge des familles. En effet, la perte d'autonomie des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées devrait être prise en charge à 100 % par la sécurité sociale et gérée par la branche assurance maladie. Selon nous, il y a véritablement urgence à créer un grand service public national de la perte d'autonomie et de l'accompagnement, incluant les établissements médico-sociaux et les aides à domicile, qui aurait vocation à revaloriser tous ces métiers

sans surprise, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 8 juillet dernier n'a pu s'accorder sur les projets de loi organique et ordinaire relatifs à la dette sociale et à l'autonomie. On peut relever deux points de divergences majeurs, l'un concernant la reprise d'un tiers de la dette hospitalière par la Cades, pour un montant de 13 milliards d'euros, et l'autre la règle d'or appliquée aux finances de la sécurité sociale. En première lecture, le Sénat a validé une grande partie de la reprise de la dette sociale par la Cades. Ce transfert nécessite une prolongation de neuf ans du versement de la CRDS pour résorber les déficits des comptes sociaux.

dont 92 milliards au titre des déficits prévisionnels des quatre ans à venir et 13 milliards de dette hospitalière. Dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, nous comprenons la prolongation de la résorption des déficits sociaux. La reprise d'un tiers de la dette hospitalière a été annoncée par l'État avant la crise sanitaire. Nous partageons

Par ailleurs, nous sommes opposés au détournement de la CRDS, dont l'existence n'a pas vocation à être pérennisée au-delà des conséquences économiques de la crise sanitaire que nous traversons. Autre point clivant, la règle d'or instaurée par le Sénat à partir de 2024 devrait permettre de garantir un solde cumulé positif ou nul sur cinq ans, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et le Fonds de solidarité vieillesse Dans la mesure où il s'agit d'un système souple autorisant les dépassements en cas de circonstances exceptionnelles, nous y sommes favorables. Il nous faut néanmoins rappeler que les efforts de maîtrise des dépenses demandés aux hôpitaux ces dernières années étaient trop importants au regard des objectifs fixés par l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam). Ce texte permet aussi d'ouvrir la voie à la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale consacrée à la perte d'autonomie et à la dépendance, que l'on La remise, fin septembre, au Parlement d'un rapport relatif à la dépendance des personnes âgées et handicapées permettra d'inscrire cette réforme dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est la consécration d'un fléchage financier spécifique C'est la consécration d'un fléchage financier spécifique de la sécurité sociale pour la dépendance. Force est de constater que les besoins financiers en la matière sont grandissants. Il faut donc les anticiper. En 2040, selon les prévisions, 14,6 % de la population aura plus de 75 ans, contre un peu plus de 9 % en 2015. Bâtir cette cinquième branche relève d'une nécessité humaine et sociale. C'est même un véritable enjeu pour nos sociétés que d'accompagner le vieillissement et la dépendance. Il s'agit d'une véritable mesure de solidarité intergénérationnelle.

texte ! En effet, la première chose que vous nous avez dite était que le Sénat avait adopté une cinquième branche de la sécurité sociale. Or, au départ, ce sujet n'avait rigoureusement rien à voir avec les textes que nous étudions aujourd'hui.

pouvait occasionner. Malheureusement, avec la crise sanitaire, la bulle a explosé et nous ne pouvions pas faire autrement que d'approuver cette pure gymnastique d'orthodoxie financière, afin de rétablir les comptes de l'Acoss. Voilà pourquoi le Sénat a suivi le Gouvernement ; c'était incontournable.

Je constate simplement que, depuis nos débats, le Ségur de la santé, qui devait trouver des solutions, tout à fait justifiées et que tout le monde attendait, concernant la revalorisation des rémunérations des soignants, qui l'avaient amplement méritée,

aurait dû être la contrepartie d'une proposition ou d'un projet de votre gouvernement, reposant sur une réforme en profondeur du système de santé. Naturellement, si vous nous aviez convaincus de la pertinence de cette réforme, nous aurions approuvé que

sur cette cinquième branche de la sécurité sociale, sur cette restructuration du système de santé, sur la règle d'or et sur l'équilibre des comptes sociaux,

Le déficit de la sécurité sociale pour 2020- plus de 50 milliards d'euros - échappe à toute référence historique. Il est accentué, rappelons-le, par l'absence de compensation, par l'État, des différentes mesures d'allégement de cotisations,

l'État emprunte à des conditions plus favorables que les agences, il gère la dette à long terme, ne supporte que les intérêts et il réemprunte continûment le principal. L'argument de la spécificité de la dette sociale n'est pas décisif, eu égard aux masses concernées, 650 milliards d'euros de dette générale. Des économistes, les organisations syndicales et le Haut Conseil du financement de la protection sociale ont ont argumenté en faveur d'une autre solution ; ce n'était pas une solution miracle, mais elle aurait libéré une dizaine de milliards d'euros de recettes sociales par an, permettant de construire un nouvel équilibre financier durable de la sécurité sociale, face aux défis nouveaux, dont ceux de l'autonomie, de de l'hôpital et des nouvelles thérapies. Au regard de cette occasion manquée, la prise en charge incongrue, par la Cades, de l'amortissement d'un tiers de la dette hospitalière, pour un coût de 13 milliards d'euros,

Le rapport Laroque, en 1962, marquait la naissance de la politique de la vieillesse ; il appelait à appréhender les problématiques de façon globale. Soixante ans plus tard, la réalité démographique impose un autre défi. L'année 2030 sera porteuse d'un symbole fort pour la première fois, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Madame la ministre, après les effets d'annonce sur ce moment historique de la sécurité sociale, la cinquième branche reste à construire. Cette branche renvoie à la place que notre société accorde aux personnes âgées ou en situation de handicap. Un financement pérenne et sanctuarisé, des prestations homogènes à l'échelle nationale, une coordination des acteurs sociaux, sanitaires et médico-sociaux sont à définir, en parallèle d'un investissement dans la prévention, du renforcement de l'attractivité des métiers du grand âge, de l'accompagnement pour les proches aidants et de moindres restes à charge dans les établissements. Le rendez-vous est donc pris.

mixte paritaire ne soit pas parvenue à un accord. Deux points d'achoppement ont conduit à cet échec : le transfert de la dette des hôpitaux à la Cades, pour 13 milliards d'euros, et la mise en place de la règle d'or, destinée à encadrer les futures lois de financement de la sécurité sociale. En ce qui concerne la prise en charge, par la Cades, de l'amortissement d'un tiers de la dette hospitalière, je rappellerai que ces dépenses visent à rembourser

déjà des mesures très fortes pour l'autonomie » et il a estimé que cette idée devait « s'insérer dans une réflexion plus large sur l'évolution du pilotage des finances sociales Je pense au contraire qu'une telle disposition, qui vise à empêcher la constitution de nouvelles dettes de la sécurité sociale, avait légitimement sa place dans ce texte. inspirée notamment des travaux du Haut Conseil du financement de la protection sociale de novembre dernier, visait à mettre en oeuvre les conditions de l'extinction de la Cades.

est, je l'ai expliqué en première lecture, particulièrement favorable à la mise en place d'une cinquième branche. Pour mémoire, en 2060, les personnes de plus de 85 ans seront près de 5 millions, contre 1,4 million aujourd'hui ; la mise en place de cette cinquième branche nous semble donc plus que jamais nécessaire.

Une réforme de cette ampleur méritait, de notre point de vue, un texte à part entière, comme cela avait été le cas, voilà vingt-six ans, avec la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. Il serait grand temps d'avoir un véritable débat sur les moyens que nous souhaitons mettre en oeuvre pour assurer la prise en charge de la perte d'autonomie et pour permettre à nos aînés de bien vieillir, de mieux vieillir. Dans quelques minutes, le rapporteur général nous présentera deux motions tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi et sur le projet de loi organique, au motif que l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, rétabli sa version sur les deux points majeurs de divergence. Si j'entends les arguments avancés, je ne peux y souscrire, car ce choix nous prive d'un nouvel examen, déjà considérablement raccourci par le recours à la procédure accélérée,

particulièrement attaché au débat entre les deux chambres, chaque fois que cela est possible, le groupe du RDSE ne soutiendra pas ces motions, qui nous empêchent de poursuivre nos délibérations.

la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant quelques mois grève lourdement les comptes sociaux de notre pays. L'augmentation des dépenses de l'assurance maladie, la détérioration de la masse salariale et les reports de paiement des cotisations et contributions sociales expliquent les prévisions les plus alarmistes. En conséquence, pour sécuriser durablement le paiement des pensions et des prestations sociales, le projet de loi ordinaire relatifs à la dette sociale et à l'autonomie prévoient un nouveau transfert de dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale vers la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

La création d'une règle d'or d'équilibre financier pour la sécurité sociale a ainsi été supprimée, les députés estimant à raison qu'une telle mesure était prématurée et que la trajectoire pluriannuelle restait à construire.

j'ai pu le souligner à plusieurs reprises, au cours des dernières semaines. D'abord, les établissements de santé sont financés en très grande partie par les caisses primaires d'assurance maladie, ce qui n'en fait donc pas une opération contre nature, comme cela a pu être avancé.

Les établissements de santé attendent avec impatience que nous fassions un geste à leur égard. Ils retrouveraient, dans cette opération financière, attendue de longue date par les professionnels de santé, une visibilité et des marges de manoeuvre qui leur font actuellement défaut. À ces 13 milliards d'euros, qui correspondent au tiers de la dette des établissements de santé, s'ajouteront les 6 milliards d'euros supplémentaires prévus dans le cadre du Ségur de la santé. Cela portera ainsi à 19 milliards d'euros l'investissement réalisé dans notre système de santé, car il s'agit bien d'un investissement,

Nous nous réjouissons en revanche du vote en faveur de la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale. Consacrée à la prise en charge de l'autonomie, cette branche offrira une ossature aux politiques existantes, facilitera la mise en oeuvre de nouvelles mesures et encouragera une approche plus préventive de la perte d'autonomie. Les précisions apportées par le Sénat ont été conservées

Ces échanges serviront à enrichir le rapport qui sera remis au Parlement, en septembre prochain, sur le financement et la gouvernance de cette nouvelle branche. Nous ne le dirons jamais assez : cette réforme ne doit pas passer à côté de la question du handicap. Les gouvernements précédents avaient esquissé les contours de la prise en charge de ce nouveau risque. Nous voici désormais à l'aube d'une réforme d'envergure, que viendront compléter, à l'automne prochain, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et un projet de loi consacré au grand âge et à l'autonomie.

Tout comme la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 8 juillet dernier, je serai brève, d'autant que je suis la dernière à intervenir dans cette discussion générale. Je serai brève, parce que les dispositifs des projets de loi ont été maintes fois rappelés. Je n'y reviendrai pas. Je serai brève encore, parce que le groupe Union Centriste, par les voix d'Olivier Henno et de Jocelyne Guidez, a déjà exprimé son sentiment, tant sur la reprise par la Cades de la « dette covid » que sur la création d'une cinquième branche. Je ne développerai que mon étonnement concernant l'échec de la commission mixte paritaire. été surprise ... Constatant l'échec de la commission mixte paritaire, son président, M. Jean-Paul Mattei, a regretté l'impossibilité de trouver un accord, car il avait bien senti que, en échange du maintien de la règle d'or, « nos amis sénateurs étaient ouverts à une reprise, même partielle, de la dette hospitalière.

madame la ministre, l'article 45 de notre Constitution est clair : le Gouvernement n'assiste pas aux commissions mixtes paritaires. Il est donc regrettable que son ombre plane sur tout particulièrement dans cette situation. S'il convient de voter des textes applicables, puisque, comme le soulignait le Premier ministre la semaine dernière, l'intendance ne suit plus,

Ainsi, son texte reprenait l'ensemble des mesures proposées par l'Assemblée nationale, alors même qu'un doute sérieux existait concernant la cinquième branche, son périmètre et son financement et sans en connaître les modalités d'application- en d'autres termes, sans savoir si l'intendance pourrait suivre ni comment. Bien que nous ne proposions que quelques ajustements de bon sens, comme le rappelait le président de la commission mixte paritaire, « le Sénat était prêt à revenir sur l'un des deux ajustements proposés. que l'a rappelé le président de notre commission, M. Alain Milon, notre souhait était d'assurer la pérennité de la sécurité sociale. En effet, notre rapporteur général, Jean-Marie Vanlerenberghe, soutenu par la majorité de la Haute Assemblée, avait fait adopter une règle d'or pour les comptes de la sécurité sociale. Cette règle se serait appuyée sur les éléments de pluriannualité qui existent déjà dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. En vertu de cette règle, le solde cumulé des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse sur les années à +4 devait être positif ou nul. Cette règle aurait été à la fois contraignante et souple. En somme, nous ne proposions qu'un décalque de ce que soutenait, à l'époque, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Olivier Véran, aujourd'hui ministre des solidarités et de la santé, pour l'examen du projet de loi instituant un L'exercice de conciliation qu'une commission mixte paritaire est censée opérer aurait peut-être pu aboutir à l'adoption d'un texte avec une règle d'or assouplie dans sa durée, par exemple, mais l'amendement de suppression déposé par le Gouvernement en séance publique au Sénat me laisse penser qu'aucune adaptation n'était vraiment autorisée.

Vouloir préserver notre pacte social nous oblige aussi à en garantir la soutenabilité dans la durée. [ ...] Ce qui révélerait une dégradation plus structurelle de nos comptes sociaux exigera des mesures de retour vers l'équilibre.

J'ai bien écouté vos différentes interventions. Je prends note, bien sûr, de votre vigilance sur la traduction dans les faits de la création de la cinquième branche. Vous savez bien que, dans le chantier que je vais mener, je serais d'autant plus vigilante que cette réforme est très importante pour moi.

Nous souscrivons évidemment à l'idée de mettre en place, à terme, une règle d'équilibre de valeur organique. Néanmoins, regardons les faits. Les prévisions font apparaître un déficit de près de 50 milliards d'euros pour 2020. L'incertitude reste grande. La trajectoire pluriannuelle reste à construire. L'adoption d'une règle d'or aussi contraignante sur un champ aussi large semblait donc trop précoce. Nous souhaitons qu'une discussion puisse avoir lieu sur une vision pluriannuelle des besoins de financement de la sécurité sociale avant de nous interroger sur l'opportunité, le sens et le périmètre d'une règle d'or. Quant à la reprise de la dette des hôpitaux, les établissements de santé sont financés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'assurance maladie. Le soutien financier à couvrir les échéances d'emprunts sera donc réalisé par celle-ci. Le Conseil d'État a souligné, dans son avis public,

de cette nouvelle lecture. Nous nous abstiendrons sur la présente motion, parce qu'elle est fondée sur le refus par la commission mixte paritaire de mettre en place une règle d'or.

sociale. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique.

des demandes d'explication de vote ? ... Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi. rappelle également que l'avis du Gouvernement est défavorable. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.